La séance est ouverte, le compte rendu analytique de La présente séance a été distribué, il n'y a pas d'observation, le procès verbal est adoptée sous les réserves d'usage. J'ai le regret, nous faire part du décès de notre ancien collègue Jean-Pierre à Philippe, qui fut sénateur de la Haute-Garonne de 1980 à 1998. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2017 adopté par l'Assemblée nationale. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des finances Monsieur le président, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général. Mesdames et messieurs les sénateurs. Si nous sommes de nouveau réunis dans votre hémicycle aujourd'hui pour une nouvelle lecture de ce 1er projet de loi de finances rectificative, c'est que le Sénat. N'a pas voté l'article 1er de ce texte en première lecture. Votre commission des finances, a voté ce matin une question préalable qui confirment l'opposition de principe du Sénat sur ce texte, je regrette cette décision, car pour ma part, je pense n'avoir jamais refusé la discussion sur ce sujet. Je suis évidemment qu'il s'agit d'une décision politique difficile. Je sais que nous demandons à nos grandes entreprises, celles qui ont plus d'un 1000000000 d'euros de chiffre d'affaires, un effort important. Mais un effort nécessaire. Nécessaire, d'abord pour garantir la bonne tenue, nos comptes publics n'aurait été beaucoup plus facile pour moi de dire, mais c'est 10 milliards d'euros. Je n'y suis pour rien. C'est la gestion précédente. Donc nous l'intégrons dans le déficit et puis nous laissons faire. ça n'est pas ma conception de la bonne tenue des comptes de la nation. J'aurais été plus facile d'aller expliquer à nos partenaires européens et bien écoutez, c'est 10 milliards d'euros, nous n'en sommes pas responsables. Nous laissons filer les déficits. Et nous ne respectant pas nos engagements européens. ça n'est pas ma conception du respect des engagements que nous devons à nos partenaires européens et à la construction européenne. Je constate d'ailleurs. Que vous avez pris la décision d'annuler cette proposition mais que personne ne m'a fourni une proposition alternative qui puisse tenir la route. Et que donc vous assumez cette idée d'avoir des déficits plus importants et le non-respect de nos engagements européens. Nous avons une exigence de rendement 5 milliards d'euros, nous avons une exigence de solidité juridique de propositions. Et nous avons enfin une exigence comptable qui est d'imputer ces 5 milliards d'euros sur l'exercice 2017, c'est-à-dire avant le 20 décembre. Il y a tous ceux qui me disent que nous allons trop vite s'ils ne l'ont pas à cette vitesse-là, ce sera demain, trop tard pour imputer ces 5 milliards d'euros à l'exercice 2017. Respecter nos engagements européens et bien tenir les comptes de la nation, monsieur le rapporteur général, je vous en suis reconnaissant que vous avez reconnu vous-même que les exigences comptables faisait que nous devions trouver 5 milliards d'euros pour 2017, le même fait des propositions sur lesquels n'ont pas pu trouver d'accord mais je reconnais bien volontiers que vous avez fait ses propositions pour que les 5 milliards soit imputée dès 2017. Je n'ai rien cacher sur. Les effets de cette contribution exceptionnelle. J'ai toujours dit qu'il y aura des gagnants et qu'il y aurait effectivement des perdants. Et j'ai toujours procédé avec la plus grande transparence. Et je vous informe que je transmettrai tous les chiffres. De cette contribution exceptionnelle dans un rapport qui sera fourni au Parlement décembre avec des chiffres complémentaires quand nous aurons l'inquiétait gravité de demandes de remboursement qui vous seront fournies dans le courant du mois de janvier. Je tiens sur cette affaire, comme sur toute la gestion des comptes publics de la nation, à ce que le Parlement soit intégralement informé et que la transparence soit au coeur de nos débats, sans quoi il n'y a pas de débat responsable possible. Je tiens à rappeler également à ceux qui considèrent que cette contribution est un juge que c'est une contribution exceptionnelle qu'elle n'a pas vocation à se renouveler et qu'elle ne se renouvellera pas. Je tiens à rappeler que les grandes orientations. Le projet de loi de finances pour 2018. Les grands augmentation fiscale du gouvernement restent les mêmes, baisser l'impôt sur les sociétés qui sera ramené de 33,3 à 25 pourcent,, mettre en place un prélèvement forfaitaire unique à 30 pourcent.. Les revenus du capital, supprimer l'impôt sur la fortune, toutes ces décisions fiscales reste inchangé et cette contribution reste une reste une contribution exceptionnelle. Je tiens enfin à ce que toutes les responsabilités soient établies. Sur cette affaire de l'annulation de la taxe à 3 pourcent sur sur les dividendes. C'est le sens du rapport que j'ai demandé à l'Inspection générale des finances et qui m'a été remis hier. L'objectif n'est pas de désigner un coupable et de se transformer en procureur. L'objectif là encore et de faire toute la lumière sur ce qui nous a amené à devoir rembourser dit milliards d'euros dans des délais extraordinairement court. Ce rapport est à votre disposition. Je vous recommande la lecture car il est passionnant. Remarquablement écrit et très précis. Ce rapport comprend notamment une chronologie très précises des sectes. Est ce qui l'établit. C'est comme au moment de la décision sur la taxe à 3 pourcent sur sur les dividendes. Personne n'a vu la difficulté. Et que ceux qui, au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale. Avait soulevé les difficultés. Il avait soulevé sur le fondement du mauvais article de la directive sur l'imposition merci. Il avait soulevé sur la base de l'article 5 qui pose la question de la retenue à la source de ce prélèvement. En s'interrogeant sur la légitimité de ce prélèvement à la source. Alors même que la Cour de justice d'Union européenne et la Commission européenne. Par la suite, devait s'intéresser à l'article IV. IV. Cette directive et à la conformité de la taxe sur les dividendes à cet article 4 de la directive de l'Union européenne qui elle porte sur l'égalité de traitement entre les sociétés au regard de cette taxe, donc en 2012, il me semble que il était impossible d'établir les responsabilités des uns ou des autres, en revanche, je vous recommande. De regarder attentivement ce qui s'est passé en 2015. Vous avez une procédure qui est engagée par la Commission européenne en février 2015. Une note de la direction de la législation fiscale qui alerte sur les risques d'annulation et sur les risques importants que cela fait peser sur les finances publiques françaises. Je vous invite à regarder l'augmentation très marquée des contentieux à la fin de l'année 2015, les entreprises voyant qu'il y a une procédure européenne, une procédure de la commission et un avis de la direction et gestion fiscale multiplie les procédures à l'encontre de l'État français, je pense qu'à partir de 2015. Il était clair. Que cette taxe était contraire au droit européen, que les risques d'annulation était réelle et la menace pour les finances publiques. Le plus important à mes yeux. C'est moins le passé. Que ce que nous en tirons comme leçon pour l'avenir. Je fais donc un certain nombre de propositions. Pour que les failles qui établit ce rapport de l'IGF. Ne se renouvelle pas par la suite et nous sommes tous concernés. Le gouvernement. Les parlementaires. C'est l'ensemble des représentants et des responsables politiques français qui je pense doivent améliorer les dispositions politiques et institutionnelles en regardant la loi fiscale. Pour garantir à nos compatriotes, la sécurité de la législation fiscale et la stabilité de la législation fiscale, c'est en tout cas les 2 objectif que je fixe : sécurité et stabilité pour notre loi fiscale dans les années à venir, je vous propose à cette fin, 3 jeux objectif. Le 1er c'est un renforcement de la sécurisation de la procédure d'élaboration de la loi fiscale parce qu'on voit bien à l'aune de cette affaire que notre procédure insatisfaisante. Incomplète et pas suffisamment rigoureuse. Nous devons prendre le temps de garantir la robustesse Riddick des dispositifs votés, nous devons davantage associer les parties prenantes, les entreprises. Les contribuables. Le Conseil d'État, la Commission européenne, toutes les parties prenantes doivent être davantage consultés pendant la procédure d'élaboration de la loi fiscale. Je vous propose en 2ème lieu davantage de transparence sur les risques de contentieux. Quand il y a une alerte de la Commission européenne. Ou de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle ne doit pas rester dans le secret de l'administration fiscale ou du gouvernement. Elle doit être transparente et les alertes plus cynique flic hâtive, je vous propose qu'elle fasse l'objet d'une information de la commission des finances de l'Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat qui disposeront ainsi toutes les informations nécessaires sur les risques de contentieux et qui en tireront les conséquences. Enfin, je vous propose 3ème objectif : une remise à plat du dispositif administratif de suivi du contentieux fiscal et la mise en place d'une procédure d'alerte plus efficace pour que lorsque nous savons que le contentieux peut déboucher les décisions nécessaires soient prises, ce qui n'a pas été le cas. Dans cette Dans cette affaire de la taxe à 3 pourcent sur sur les dividendes. Je souhaite que nous engagions ce travail sur la base de ces objectifs. Je vous propose que Sénat-Assemblée nationale gouvernement travaillent ensemble sur la base de ces objectifs et des autres propositions qui sont faites par l'IGF sur l'amélioration de la le bar ration de la loi fiscale j'y attache une importance considérable. Je considère que ce qui s'est passé une fois et qui menace nos finances publiques qui menace le respect de nos engagements européens ne doit pas se renouveler une 2ème fois et qu'il n'y a qu'en allant au fond du sujet. En traitant les problèmes à la racine que nous remet diront aux failles de la Logan ration de la loi fiscale français voyez propositions que je voulais vous faire aujourd'hui en profitant de notre discussion, tout cela est évidemment ouvert à discussion devant vous, je souhaite que nous puissions continuer à échanger sur ce sujet, nous aurons d'autres occasions pour parler plus globalement du PLF 2018, je serai devant vous la semaine prochaine pour défend devant vous la transformation en profondeur de la fiscalité, telle qu'elle est proposée par le gouvernement aujourd'hui, le sujet n'est pas là, il s'agit de tourner la page de cette taxe, arrivé à financer le manque à gagner pour l'État et le respect de nos engagements européens, telle est aujourd'hui l'objet d'autre débat je vous remercie. Si la parole est à monsieur Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre prend la commission des finances, mes chers collègues, le conseil des ministres examinera demain le vrai collectif budgétaire, si je puis dire, celui de fin d'année qui procède aux ajustements nécessaires traditionnellement à la fin de l'année et nous sommes amenés à revenir cet après-midi sur ce collectif budgétaire d'urgence sur ce sujet que nous connaissons bien, puisque, comme vous savez, s'était dit à l'instant, la commission mixte paritaire ne n'a pas abouti, n'a pas abouti puisque le texte qui nous occupe aujourd'hui comportez vous le savez, 6 articles à l'issue de la discussion, en première lecture par la sur les nationales, le Sénat en adopté 4 conformes ne sont pas les plus importants et, évidemment, on a modifié 2 et d'où l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie vendredi dernier, vous savez que notre divergence, elle porte sur un point essentiel, c'est l'article 1er du projet de loi, l'article 3 l'autre article non adopté mais évidemment que la de quoi s'agit-il, par le gouvernement parlait, c'était de faire face au remboursement de la taxe validé sans pour autant compromettre le retour aux 3 pourcent donc donc l'objectif de sortie de la France de la procédure de déficit excessif en 2017, néanmoins le Sénat évidemment regarder l'incidence de cette taxe qui touche particulièrement certains secteurs, je pense au commerce, je pense aux services financiers et notamment aux banques mutualistes c'est incidence a été très largement souligné lors de débats, de même que être et souligné le message quelque peu contradictoire entre la baisse annoncée dans le PLF de l'impôt sur les sociétés et cette surtaxe certes exceptionnel, c'est la raison pour laquelle le Sénat a donc supprimé, c'est des surtaxes, bien entendu, on ne peut lectures le l'Assemblée nationale a souhaité revenir à ce texte de premières lectures, il y a une petite correction sur l'article 1er de rédactionnel et d'un sous-amendement du garnement sous- amendement qui supprime dans le rapport, qui va être présenté au Parlement, la mention des entreprises perdantes et gagnantes, ça sera remplacée par une présentation plus large à l'échelle de la société ou d'un groupe de sociétés,

nous avons donc à cette période d'une certaine mais manières une connaissance précise de l'impact de ces mesures fiscales après l'adoption de celle-ci, la somme les national enfin adopté pour être complet, l'article 3 dans sa rédaction telle qu'elle est issue des travaux de premières lectures, alors pourquoi une question préalable, je n'ai pas mis à étendre longuement, nous avons eu un long débat avec différentes positions qui sont exprimées la semaine dernière nous sommes manifestement de la possibilité de rapprocher les positions que je peux été exprimée d'une part par l'Assemblée et, d'autre part, par le Sénat et qui s'est désaccord a été évidemment marqué en commission mixte paritaire, c'est la raison pour laquelle la commission des finances, considérant que le débat a eu lieu, c'est pas pour autant en approuver ou désapprouver la position du garnement nous considérons simplement que ce débat est largement lieu et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir et que les positions exprimées par les 2 assemblées sont irréconciliables et c'est la raison de cette question préalable sur ce projet de loi de finances rectificative, donc je pense que nous partageons tous, surtout le banc sans doute une opinion égal il est temps de sortir de ce débat qui appartient sans doute peut-être passé j'espère demain parlé des conclusions de de la l'Inspection générale des finances pour moi ce qui m'intéresse, c'est moi la partie sur le passé est le passé, le passé et il a fait à l'instant même quelques propositions qui auquel je je ne peux souscrire, notamment celle de mieux anticiper de mieux préparer la loi de finances, celle également d'être mieux informés, il y a une proposition très précise du rapport de l'IGF sur la sur la formation des présidents et rapporteurs généraux sur les risques contentieux nous y souscrivons et nous sommes tout à fait prêt Monsieur le ministre, à travailler pour que la loi soit mieux préparé et qu'à l'avenir

alerté le gouvernement de l'époque sur les risques constitutionnels, nous n'avions pas été entendus, donc nous aurons à prendre mieux en compte ces risques comptables communautaire et constitutionnel, à l'avenir, alors simplement Monsieur ministre était une demande, c'est que ce que vous formulez aujourd'hui comme une bonne intention à laquelle on souscrit ne vaille pas simplement pour les PLF mais également pour les PLFR les faire parce que l'expérience prouve que pour les collectif budgétaire de fin d'année, nous avons parfois en séance parfois très tardivement dans la précipitation des amendements parfois technique parfois beaucoup moins technique mais plus politique qui nous parviennent, avec parfois une absence totale ou quasi totale d'expertise juridique et le Conseil constitutionnel est régulièrement amené à statuer, soit par des QPC soit par une saisine initiale et annulé ces dispositions comme la précipitation et le bricolage fiscal malheureusement donne des mauvais résultats et c'est peut-être l'enseignement dont nous devons tirer pour sortir peut-être positivement de mauvaise passe merci et j'espère que

Merci, monsieur le rapporteur général dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Julien Bargeton. Pour 6 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des finances Monsieur, rapporteur général mais, chers collègues, les séances se suivent et, hélas, cela se ressemblent, lecture et nouvelle mais le débat, l'est moins, c'est de bonne guerre, n'y voyez pas là le signe d'un spleen baudelairien de l'Automne, mais plutôt une réelle déception à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire de vendredi dernier, car monsieur rapporteur générale cher que l'aide de la majorité sénatoriale, nous aurions pu nous mettre d'accord sur ce texte vous en avait décidé autrement en 6 minutes chrono, je le regrette car ce texte est un texte grave, le gouvernement a su tirer les conséquences budgétaires de la décision du Conseil constitutionnel, rendu le 6 octobre pas de dilution, pas de jeu de cache-cache la sincérité, ce collectif budgétaire n'est pas qu'une affaire de chiffres, il est une affaire de souveraineté la crédibilité budgétaire de notre pays et la condition sine qua none du retour de la France en Europe depuis 2009 et des majorités se sont succédé, la France est en procédure pour déficit excessif, avec ce texte proposé par le gouvernement, nous avions une occasion de sortir par le haut de cette épreuve en sécurisant notre trajectoire de finances publiques, vous en avait décidé autrement, chers collègues de la majorité sénatoriale, vous auriez pu prendre des gants, vous avez préféré rejeter tout de Go la rédaction de l'article 1er instituant 2 contributions exceptionnelles à l'imposition sur les sociétés, je ne reviens pas sur le dispositif, mais je rappelle que le gouvernement s'est efforcé de concentrer ses contributions sur les plus grandes entreprises bénéficiaires, et j'insiste à dessein sur ce mot bénéficiaires, c'est le principe même de l'impôt sur les sociétés, il ne faut donc pas dire que l'ensemble des entreprises et même l'ensemble des grandes entreprises seront taxés comme dans tout dispositif fiscal il y a des gagnants et des perdants entre ceux qui seront remboursées au titre de de la taxe sur les dividendes et ceux qui devront s'acquitter dans quelques semaines de la contribution exceptionnelle, mais c'est évidemment habituel et le gouvernement, et d'ailleurs c'est aussi entre Rhodes de Transe de parlementaires veillera à les effets de aux effets transfert, cela a été dit, vous avez préféré donc un texte déséquilibré qui penche beaucoup avec la dépense de remboursement, mais sans la recette, c'est paradoxal pour les thuriféraires déséquilibres publics, ce n'est pas parce qu'il y a une Exposition consacrée à René Goscinny en ce moment à Paris que je vous invite à aller voir, mais le texte du Sénat ressembler un peu aux constructions de Numérobis seul architecte de Cléopâtre, vous savez qui a été un peu bancal ne il ne suffit pas de de dénoncer les les trains en retard, les déraillements à venir mais il ne faut pas non plus laisser les Français sur une voie de garage, comment qualifier autrement, une attitude qui consiste à supprimer un dispositif qui permet à notre pays de respecter les engagements comment expliquer à nos concitoyens qu'il est finalement urgent d'attendre, comment justifier cette décision devant nos partenaires européens, je ne peux pas croire que vous ne partagez pas mon jugement Monsieur rapporteur général une impasse budgétaire est une impasse politique, c'est une impasse démocratique, un texte d'urgence n'est pas le véhicule juridique approprié pour revoir les hypothèses de croissance, sauf à vouloir faire passer un chameau par le trou d'unique, je suis convaincu que nous parviendrons à travailler de nouveau de manière intelligente et constructive, une fois le mois de décembre passé vivement décembre si j'ose dire, la première partie du PLF 2018 que nous allons examiner demain en commission comporte des mesures extrêmement positive est attendu en faveur du pouvoir d'achat des ménages et de la compétitivité des entreprises, j'ignore à quoi il faut s'attendre de la part de la majorité sénatoriale, mais j'espère une attitude responsable, une attitude constructive plutôt que cette fois, un rejet du l'état d'esprit du groupe, la République en marche est quant à lui, résolument en tournée vers l'avenir, nous devons collectivement nous poser la question : comment mieux travailler, nous parlementaires vous gouvernement pour éviter ce genre d'OFNI, objet fiscal non d'identifier, je l'avais indiqué jeudi soir mais ma position est constante, je suis favorable à la mise en place de nouveaux outils de contrôle du suivi des contentieux fiscaux au Parlement, c'est d'ailleurs la partie la plus intéressante du rapport de l'IGF qui, elle, a été remis sur cette triste histoire, la sécurisation de la l'élaboration de la loi fiscale, nous avons le devoir de bien veiller à la bonne gestion des deniers publics par le gouvernement et cet cet épisode ne fait que renforcer cette exigence les censure du Conseil constitutionnel ne sont que le reflet de nos insuffisances collectives, il faut donc mieux prendre le temps de l'évaluation, plutôt que de céder, comme c'est parfois le cas à l'emballement, il y a la précipitation, Monsieur le Ministre, vous avez formulé des propositions, et là encore, je ne doute pas de la bonne volonté de de la majorité sénatoriale de tous les groupes pour les regarder avec attention pour résumer et sans naïveté aucune cette nouvelle lecture aurait dû être une invitation à renouer le dialogue, cela aurait été une belle image de notre assemblée, donner à nos concitoyens, leur montrer qu'au-delà de nos parcours et couleur politique, nous savons aussi nous rassembler sur dans les moments difficiles, la question préalable est l'ultime illustration de sa tête attitude d'obstruction qui n'est pas à la hauteur des enjeux du texte, à défaut de vous convaincre, je la regrette, sans préjuger des débats plus fructueux, à l'avenir, notamment sur les sujets de fond que vous avez abordé, monsieur le Ministre, en matière d'élaboration de la loi fiscale, je vous remercie. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Un petit mot trivial, mais j'ai l'impression groupe on a l'impression qu'il ne qui dispute des droites. Donc c'est un fait. Pour 2 raisons essentielles sont de nature politique et on peut les comprendre, vous êtes d'accord. Sur les contraintes qu'ont été celle du traité voté il y a 5 ans, et où les appliquer. Et deuxièmement, quand il s'agit de voter la baisse de la dépense publique, vous la voter ensemble. Que ça soit l'Assemblée ou presque au Sénat.

Et je suis pas dans le passé, qui avons rapporté 15 milliards à l'État. C'est intéressant quand même. C'est l'entreprise Orange. L'opérateur historique du téléphone à durant l'année 2016 génère un chiffre d'affaires de 23,5 milliards d'euros environ. L'excédent brut d'exploitation de l'entreprise est proche de 4 milliards et sa politique de distribution de dividendes l'amener accordé près de 1,6 milliards d'euros à ses actionnaires, à ce titre-. Eh bien en 2016 catastrophe. Orange et ça a été obligé de payer 200 millions d'euros d'impôt sur les sociétés. Et j'ai, je suis rapporteur pour la commission des finances remboursements et dégrèvements. Ils n'ont même pas payé ces 200 millions en fin de compte, donc voyez la surtaxe de l'impôt sur les sociétés, elle pouvait se concevoir, mais à la quand même quelques défauts et sa portée est limitée quand même puisque je fais un calcul mais si d'autres collègues vous diront le contraire, ça fait 0 2 pourcent PIB l'envoyé personnel, monopole de l'entreprise, on pourrait prendre d'autres exemples. Mais parlons de l'entreprise, y compris au Sénat. En donnant la réalité en dans la 2ème chose c'est parce que on nous dit : on a oublié, on voulait, on peut dire que c'est une bonne intention pouvait laisser passer le contentieux de la contribution sociale bénéfice causé le bénéfice de les creuser le déficit de l'État, vous allez dire le le groupe communiste citoyens écologistes irresponsable. Franchement Crouzet, le déficit de l'État. L'État c'est nous, l'État, c'est les collectivités, l'État, c'est des citoyens. Mais nous, on avait preuve de responsabilité, puisque nous l'avons fait dans les amendements que ça soit l'Assemblée où le groupe respectif et ici au Sénat. C'est que ça pouvait certes creusé le déficit de l'État mais là serait une irresponsabilité si on n'avait pas été chercher d'autres recettes. On nous dit ça va pas du tout, c'est la catastrophe. Vous me dites si je me trompe. Jeanne devoir que France Trésor a émis il y a un mois, donc on est, on est vraiment dans la conjoncture actuelle. 4371 millions d'obligations de moyens termes à taux 0. 0. C'est pas quand même la grande catastrophe des comptes publics et puis si on voulait pas avoir les désagréments qu'on a là, y compris avec le respect, on peut avoir de l'État. Ou s'acheter des mots à la figure, pour faire des fausses disputes ou inventer fausses divergences quant on est d'accord. Il y avait un truc qui était très mais collègues. Il y a pas de problèmes techniques, il y a pas de problème juridique. Il fallait prolonger la majoration de l'impôt sur la solidarité. Et là, on n'aura pas de problème, on n'aurait pas eu la navette on vrai besoin de réunir la commission mixte et on n'avait pas de problèmes juridiques et on n'a pas de problèmes administratifs, donc on prendrait pour toutes ces raisons-là non groupe ne participera pas, ne votera pas c'est jeu collectif rectificatif budgétaire. Vous avez vu, j'étais sérieux en nombre de minutes et merci de votre attention. La parole est à monsieur Bernard Delcros pour 8 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, la commission des finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues, vendredi, la commission mixte paritaire s'est soldée par des chèques, ça n'est pas une surprise, c'était prévisible nous examinons donc en nouvelle lecture, comme cela a été dit au lendemain du vote de l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances rectificatif pour 2017 alors que ce ressortir de nos débats de la semaine dernière en première lecture une majorité finalement s'est dégagée au Sénat pour supprimer l'article 1er à l'issue d'un scrutin public et ce. Malheureusement, sans proposition alternative permettant de tenir nos objectifs budgétaires et nos engagements européens, pour notre part, nous le regrettons. D'autant que tous les amendements déposés sur l'article 1er avait préalablement été rejetée y compris un amendement de suppression de l'article. En réalité, l'article 1er est au coeur même du projet de loi celui qui instaure la taxe exceptionnelle sur les sociétés dont je le rappelle, le chiffre d'affaires est quand même supérieur à un 1000000000 d'euros en plus avec une progressivité contribution exceptionnelle que le gouvernement veut mettre en place pour faire face au mieux aux conséquences financières de la censure par le Conseil constitutionnel de la taxe sur les dividendes, créée en 2012. Et bien sûr, ce rejet pur et simple de l'article 1er a eu pour effet de supprimer les 2 contributions, nous avons dû tirer les conséquences de cette décision. Avec un amendement présenté par le gouvernement dans la foulée pour procéder à l'ajustement de l'équilibre financier pour cette perte de 5,4 milliards d'euros de recettes. Par voie de conséquence, le déficit budgétaire de l'État, tels qu'ils résultent et la délibération du Sénat ressortait à 88 7 milliards d'euros à la place des 76,9 milliards d'euros prévus, soit une dégradation de notre déficit de 4,8 milliards d'euros. Le Sénat ayant supprimé le coeur de ce projet de loi de finances, hé bien, la commission mixte paritaire n'a eu qu'à constater l'impossibilité d'un accord entre les 2 chambres et sans surprise, après l'échec de la CNP, l'Assemblée nationale a rectifié et re-rétabli l'article 1er en nouvelle de lecture alors quelle est la situation aujourd'hui, nous sommes face à une obligation, une obligation à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire celle de rembourser 10 milliards d'euros aux entreprises taxées sur les montants distribués depuis 2013 voilà quel est concrètement la situation et voilà qu'elle est, à notre avis, la situation à laquelle nous devons répondre à responsabilité le contenu du dispositif proposé par le gouvernement est aujourd'hui bien connue, couvrir la moitié de la somme par cette imposition progressif sur les bénéfices et l'autre moitié sur un prélèvement sur le budget de l'État, alors il ne s'agit pas de savoir si la solution proposée est idéal, il n'y a pas de solution idéale, il s'agit de savoir si on a une meilleure et si oui, quelle est-elle, quelle autre solution avant nous taxer tous les Français, creuser les déficits, laisser filer l'endettement au moins bien qu'aucune de ces solutions n'est crédible au regard de la situation de notre pays. Alors qu'il ne reste plus que 3 pays sous le coup de la procédure pour endettement successives dans l'Union européenne dans la France depuis maintenant 8 ans serait irresponsable mais, chers collègues de creuser encore le déficit public de notre pays, Que nous avons par ailleurs voulu ne devons-nous pas tout faire pour alléger une dette insoutenable pour notre société et pour la France de demain. On peut dire 5 milliards d'euros supplémentaires, ce n'est pas grand-chose au regard de notre dette, et c'est vrai, mais c'est justement c'est justement en choisissant toujours cette solution-là qui consiste à dire qu'après tout ce n'est pas grand chose que notre dette frôle aujourd'hui 100 pourcent du du PIB avec 2200 milliards d'euros, ce texte au-delà de ce qu'il contient est une occasion d'agir en responsabilité, nous devons le faire au nom des générations qui viennent. C'est pourquoi, au bout, au nom du groupe de l'Union centriste nous voulons affirmer cette quand diction et c'est aussi pour cela que nous avons soutenu à l'unanimité le texte présenté par le gouvernement la semaine dernière, je rappelle que la solution qui est inscrit dans ce projet de loi ne dégrade pas notre déficit en 2017 et le creuse légèrement en 2018, je vis de 0,2 point du PIB, sans toutefois remettre en cause nos engagements européens. Certes, nous aurions tous je préférais ne pas avoir à gérer cette situation et à prendre une telle décision mais quand on l'a dit cela, on n'a rien fait, a lancé et on n'a pas apporté le moins début de solution je considère pour ma part, Monsieur le Ministre, que vous apporter une réponse pragmatique et réaliste, nous pensons que le Sénat dans sa sagesse, peut encore faire preuve de responsabilité art examinant sa position, c'est pour cela que, au groupe de l'Union centriste, à l'unanimité, nous voterons contre la motion tendant à opposer la question préalable, je vous remercie. Merci, la parole est à monsieur Claude rénal. Pour 10 minutes. Monsieur Monsieur le président, Monsieur le Ministre, monsieur le président de la Commission, monsieur le rapporteur général mis chers collègues, je ne reviendrai pas ici sur les origines de ce projet de loi rectificative ni sur les raisons de l'abstention de notre groupe en 1ère lecture me bornant renvoyé à notre débat en discussion générale de la semaine dernière, je note cependant que, depuis jeudi, le rapport de l'Inspection générale des finances que vous aviez commandé, monsieur le Ministre, amène, celle-ci a, je cite, vouloir sécuriser la loi fiscale et à vouloir sécuriser le contribuable, ainsi qu'à faire quelques préconisations en ce sens, la lecture de ce rapport, Monsieur le Ministre, nous amène bien loin du scandale d'État, voire même de l'amateurisme stigmatisés, je vous rappelle, et les quelques difficultés que nous avons pointé lors du dernier débat des entreprises de nouvelles touché par la surtaxe sur l'impôt sur le revenu notamment celles que il ya distribuent pas de dividendes, une lycéenne de gagnants et de perdants, vous l'avez dit, monsieur le ministre, non documenté à ce jour, mais des solutions alternatives, j'entends mes collègues avant moi dire il n'y a pas de solution alternative mais si, et on a proposé des solutions alternatives, le groupe communiste la proposé, nous en avons proposé notamment le report des mesures sur l'ISF ou le prélèvement forfaitaire unique, il suffisait de les reporter d'un an ou 2 pour que les choses puissent finalement ce financier, donc des solutions alternatives existent, il ne faut pas le nier, qui, en tant que telle, aurait dû, dès la première lecture nous conduire à nous opposer directement, nous avons préféré donner une chance à un accord au Sénat en nous abstenant, ce qui est un signal tout en marquant notre désaccord avec l'article 5 qui ratifie le décret d'avance du 20 juillet 2017, je dois vous dire Monsieur le Ministre, que si malgré les réserves que je viens de formuler le calendrier faisait que l'intérêt de notre pays, Apple a un vote immédiat notre groupe aurait sans doute fait l'effort nécessaire que le groupe LR par son vote négatif s'est refusé à faire, l'Assemblée nationale étant convoqué ce soir en lecture définitive, nous en resterons à notre position initiale ne pouvant dans ce projet de loi validé des dispositions très largement critiqué par notre groupe et, au-delà, ayant fait l'objet du décret d'avance du 20 juillet 2017, notamment celles concernant la baisse des APL, la suppression des contrats aidés ou la diminution de certaines aides aux collectivités concernant la question préalable par principe, je dis bien, par principe, nous ne la voterons pas, ne la jamais car elle est pour nous la négation du travail parlementaire, je vous remercie. mesure. La parole est à monsieur Emmanuel Capus pour 6 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous examinons donc à nouveau le projet de loi de finances rectificative pour 2017, le groupe les indépendants républiques et territoires défend en la matière une approche de responsabilité devant une situation impérieuses d'intérêt général. L'héritage d'insincérité budgétaire et de laxisme du précédent gouvernement menace de dégrader le solde budgétaire de l'année et de sérieusement compromettre notre sortie de la procédure pour déficit excessif dans cette urgence, nous partageons la volonté du gouvernement et du président de mettre fin le plus tôt possible à cette procédure. Nous estimons que là se trouve l'intérêt national, nous estimons que Sud c'est une condition nécessaire à la restauration du crédit de la France en Europe, nous admettons enfin que dans cette situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles sont nécessaires pour respecter nos engagements pour toutes ces raisons, nous nous opposons pas à ce texte présenté en l'état, ce projet de loi de finances rectificative néanmoins loin de répondre à l'idéal de justice que nous défendons, vous le savez, non content de faire payer aux entreprises, les erreurs de l'état, ce projet de loi pénalise les entreprises qui investissent et créent des emplois. Il crée des gagnants et des perdants sans rapport avec les politiques de distribution des entreprises sans lien avec leur Exposition à la taxe à 3 pourcent sans sans mesure enfin de leur situation financière, sur le long terme, c'est la raison pour laquelle nous déplorons que le gouvernement n'ait pas pu proposer une mesure plus fine qui répartissent plus justement l'effort entre les entreprises. Néanmoins, vous, héritez, Monsieur le Ministre, d'une situation budgétaire critique, nous le comprenons dans cette optique, dans cette optique de responsabilité, nous ne nous opposons pas à cette mesure urgente et nécessaire à la restauration de notre crédibilité en Europe. J'aurais aimé que cette nouvelle lecture soit l'occasion d'une prise de conscience, si nous échouons à sortir de la procédure pour déficit excessif en 2018, il se peut que cet échec hypothèque l'ensemble du quinquennat avec les incertitudes pesant sur l'année 2019, cela nous ne pouvons pas l'accepter. Il nous faut collectivement solder une fois pour toutes l'héritage de la crise et les errements budgétaires du passé pour enfin nous tourner vers l'avenir. Sachez néanmoins, Monsieur le Ministre, que l'indulgence de la représentation nationale s'accompagnera d'une vigilance accrue pour le futur, le nom, donc le processus d'élaboration de la loi fiscale souhaite améliorer en profondeur tout au long de la chaîne législative, vous l'avez compris : sécurité, stabilité, avez-vous indiqué, Monsieur le Ministre, nous vous en donnons acte et nous partageons ces objectifs, nous demandons que cette malheureuse affaire soit pour vous et vos services, l'occasion d'une réflexion sérieuse sur leur manière d'élaborer la norme fiscale nous demandons enfin que des mécanismes d'alerte performant soit mises en place, il faut à l'avenir, empêcher que des annulations contentieuses de cette importance ne Vienne mettre en péril la trajectoire budgétaire de la nation. Nous devons avoir conscience que nos concitoyens ne nous pardonneront pas les remèdes superficielle les expédients qui ne traitent pas les causes du mal, le précédent gouvernement a épuisé leur patience les limites du consentement à l'impôt, ont été atteints cette nième rustine doit mettre un point final à cette période d'irresponsabilité et ouvrir enfin la période de courage et de sincérité budgétaire que le président de la République nous a promis la période de sécurité et de stabilité que vous nous proposez, Monsieur le Ministre, je vous remercie. Merci, la parole est à monsieur Yvon Collin. Monsieur Monsieur le président, Monsieur le ministre. Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, comme le rappelait mes prédécesseurs, après l'échec de la commission mixte paritaire la semaine dernière, nous sommes donc amenés à examiner ce projet de loi de finances ce rectificatif pour 2017 jeudi dernier après des débats prolongés, la haute assemblée a rejeté en première lecture la principale mesure du Texas, avoir l'aime pas exceptionnel sur les grandes entreprises, je regrette, comme l'une femme de mon groupe car le refus de cette contribution signifierait s'il était adopté, le passager du déficit public de 2 9 pourcent à à 3,1 alors que la France est un des derniers états de la zone Euro, soumis à la procédure de déficit public excessif, des finances rectificative, cela est expliqué prévoit la création pour l'exercice 2017 d'une contribution exceptionnelle à l'impôt sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés de plus d'un 1000000000 d'euros de chiffre d'affaires, ainsi qu'une contribution additionnelle sur les sociétés pour les sociétés de plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est une réponse législative Mali dation par le Conseil constitutionnel le 6 octobre dernier de la taxe additionnelle de 3 pourcent sur sur les dividendes, instituée par la haute finance rectificative de l'été 2012 décision fondée je cite sur la différence de traitement entre les sociétés mères selon les dividendes qu'elles distribuent proviennent ou non de filiales établies dans les zones États-membres de l'Union européenne autres que la France le 17 mai dernier, la Cour de justice de l'Union européenne avait d'ores et déjà jugé la contribution de 3 pourcent sur sur les revenus distribués incompatible avec le régime fiscal européen commun applicable applicables aux sociétés mères filiale à la suite de ces décisions, l'État est donc tenu de rembourser les sommes perçues aux entreprises concernées, soit près de 10 milliards d'euros, un montant important, qui comprend notamment des intérêts moratoires de 4,8 pourcent par par an qui s'ajoutent leur l'aura compris, au remboursement des sommes perçues depuis 2012, je note d'ailleurs que le taux des intérêts moratoires devraient être réduit de moitié dans le prochaine avait fait rectificatif pour le rapprocher des taux d'intérêt actuel, d'après les estimations données par le gouvernement, ces dispositions concerneront environ 300000 entreprises au total donc samedi assujettis autour de 30 le rendement étant estimée à 5,4 milliards d'euros, donc 4,8 milliards d'euros versés en 2017 au titre d'un acompte payé avant le 20 décembre de cette année, 2 sortes de public 2017 serait inchangé par rapport à l'estimation réalisée lors du dépôt du projet de vote final seul pour 2000 du 18 à 2,9 au-delà de 2017 le coûte au contentieux serait intégrée à la trajectoire des finances publiques, sans compromettre pour cela le respect par la France de ses engagements européens, la prévision du solde pour 2018 prévues dans le PLF à 2 6 pourcent serait serait évaluée à 2,8 pourcent.. Le rapport de l'Inspection générale des finances remis hier au ministre de l'Économie et des Finances ministre l'a rappelé à établi la chronologie de l'adoption de la taxe sur les dividendes 200 même, tiens et en fait de son annulation cette taxe était née de la volonté de couvrir notre contentieux sur les Opcvm et de la mise en oeuvre des engagements de campagne de l'ancien président de la République sa constitutionnalité et ça comptabilité comme Patty milité avec le droit européen n'avait pas était mise en cause par l'administration, ni par le Conseil d'État, ni par les parlementaires, auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi de 2012, en revanche, les si y a des comptabilités avec le droit européen était apparu en 2015 avec une question préjudicielle sur la taxe belge similaire, mais surtout après la mise en demeure de la France par la Commission européenne sur l'incompatibilité avec la directive mères- filles sur les principes de liberté d'établissements et de circulation des capitaux et ne fait qu'avec la multiplication des contentieux à partir de cette même année, le rapport tire des leçons importantes pour l'avenir d'abord renforcer la solidité de la loi fiscale à l'image de bonnes pratiques existant dans notre pays européens, en associant davantage les acteurs publics dans le Parlement et les acteurs privés ensuite améliorer la transparence sur les risques de contentieux redéfinir en fait le suivi administratif du contentieux fiscal et mettre en place une procédure d'alerte efficace concernant le présent projet de loi la position du groupe RDSE reste identique à celle exprimée en première lecture, si le dispositif n'apparaît pas satisfaisant regard du calendrier de la méthode qu'il faudra nécessairement ça été dit, répété les des gagnants et des perdants et à plus long terme, au regard du projet du gouvernement de renforcer l'attractivité de la fiscalité des entreprises, nous pensons qu'il n'y a pas de solution alternative qui n'aurait lourdement pénalisé les finances publiques, rappelons également que l'État prend à sa charge la société pas moins de 5 milliards d'euros, soit environ la moitié du remboursement de la taxe sur les dividendes, c'est pourquoi nous ne pourrons suivre la position du rapporteur sur la motion tendant à adopter la question préalables majoritairement favorable à l'examen et à l'adoption du texte du gouvernement nous voterons donc contre cette mention, monsieur le rapporteur général, je vous remercie chaque relais. La parole est à monsieur Jean-François Husson pour 10 minutes. Monsieur

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général mais chers collègues l'Inspection générale des finances a donc rendu son rapport hier et ses conclusions sont sans appel la taxation d'entreprises. Pour rembourser d'autres entreprises, d'une taxe illégale au motif que l'urgence ne permettait pas de trouver d'autres solutions ne tient plus. L'IGF confirme ce que j'avais dit en première lecture. Le problème était identifié depuis longtemps. Et le choix du gouvernement a toujours consisté à repousser la décision, en misant sur la probabilité d'une issue d'un dénouement qui ne lui soit pas trop défavorable. Aller plus loin et plus vite dans les économies pour dégager des marges de manoeuvre. Par exemple en réduisant la dépense publique ou même vendre des participations de l'État, des solutions existaient bel et bien je rappelle que les participations de l'État, c'est aujourd'hui 100 milliards d'euros. Comme je l'avais indiqué en première lecture, Emmanuel Macron était à Bercy, à la tête du ministère de l'économie quand, en 2015 le risque a été clairement identifié pointé et signalé par le secrétaire d'État au Budget. L'Inspection générale des finances retient d'ailleurs également cette date dénonçant et je la cite le choix politique fait à partir de 2015 de maintenir la taxe est de continuer à l'apercevoir en dépit d'incertitudes adhérer sur sa conformité au droit européen. En effet, la mise en demeure par la Commission européenne en 2015 aurait dû constituer une alerte suffisante pour faire réagir Emmanuel Macron. Et Michel Sapin, alors à la tête de Bercy, d'ailleurs, si le gouvernement avait réagi fin 2015 le coup n'aurait pas dépassé les 3 milliards d'euros. Le recours devant le Conseil d'État en 2016 laisser subsister moins de doutes encore notre rapporteur général l'avait d'ailleurs clairement te évoqués, et notamment le problème constitutionnel. Alors, le gouvernement refuse de prendre à sa charge la totalité du remboursement, la fameuse somme de 10 milliards d'euros qu'il considère comme trop importante risquant en effet d'obérer la baisse du déficit public pour passer sous la barre des 3 pourcent mais j'ai à cet instant une question à formuler. La taxe sur les revenus distribués a rapporté au budget de l'État chaque année depuis 2013. 2 milliards d'euros de recettes, elle a donc malgré son caractère aujourd'hui illégale. Contribuer. à amoindrir le déficit public. Un déficit public qui calculé sur les bases corriger. Aujourd'hui devrait donc être en 2017 n'ont pas de 2,9 mais de 3,3 pourcent.. Voilà la réalité. Dont vous n'êtes pas responsable, mais vous êtes aujourd'hui comptable monsieur le Ministre, et ce sont des arguments objectifs que je veux livrer à notre assemblée. Il faut également intégrer le fait que l'économie, pour une part repose sur de la psychologie et pour le moment. Je dois avouer et je m'en réjouis que le président de la République bénéficie d'une relative bienveillance elle elle là que la confiance revient progressivement les investissements reprennent. Les embauches ont cédé et augmente, mais cette confiance. Et reste fragile, c'est la raison pour laquelle il est besoin de donner des gages, parce que les acteurs économiques ont besoin de stabilité et de lisibilité et de confiance. Pourtant, les principales mesures qui leur avait été promise pendant la dernière campagne électorale, ont déjà été repoussées à 2019. Puisqu'il n'y aura pas d'amélioration sensible attendre dans ce projet de loi de finances pour l'année 2018. Ajoutez à cela que toute erreur commise par l'État. Selon ce que vous nous proposez aujourd'hui doit être payé sur le dos et par les entreprises, c'est, je le crois, maître dangereusement en péril le lien de confiance que j'évoquais tout à l'heure. le gouvernement promet de baisser l'impôt sur les sociétés pour le ramener en 2022 à 25 pourcent.. Et voilà qu'ils commencent par augmenter ce fameux impôt pour certaines grandes entreprises, en le portant à un niveau record, qui peut atteindre 43,33 pourcent,, excusez du peu. Prendre les autres grandes entreprises ainsi en otage ou pour des vaches à lait, c'est parfois oublier que ces fleurons de notre économie sont aussi de formidables pourvoyeurs d'emplois, des milliers d'emplois et qu'elle génère également beaucoup de sous-traitance. Auprès d'autres entreprises. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que 318 entreprises seraient concernées, dont 109. Pour une une contribution dite additionnelle. 223 serait perdante, c'est-à-dire qu'elle paierait plus de surtaxe qu'elle ne recevrait de remboursement. Un tiers d'entre elles, de 2 de ses 223 serait d'ailleurs. c'est ainsi que vous le dites, c'est-à-dire que, elle, n'aurait aucun remboursement alors elle serait prélevée mais surtout. Il y a 15 jours, il n'était même pas question que ça. Ce Ce sont d'ailleurs ces entreprises bien souvent des ETI, vous savez, les fameuses entreprises de taille intermédiaire, celles qui sont les premières pourvoyeuses de création d'emplois en France, les entreprises de ta intermédiaire, celle-là même qui hante réinvesti leurs bénéfices dans la croissance plutôt que dans la rémunération d'actionnaires qui sont des entreprises ou des groupes de protection sociale ou bancaire mutualiste. Ces dernières sont impactés, un niveau record, ce qui doit nous interpeller. Ainsi, avec près de 800 millions d'euros de contributions. Dont elle n'avait pas connaissance, je le redis, il y a un peu plus de 15 jours c'est aujourd'hui plus de 15 pourcent de de la facture à la seule charge par exemple de 3 grands groupes mutualistes et coopératifs. Alors, vous parlez de perdants nets de perdants et de gagnants, je ne poserais qu'une seule question : il y a-t-il réellement des gagnants, hé bien je n'en vois pas. Les entreprises qui ont été soumises à la taxe de 3 pourcent sur sur les dividendes ont été mis à contribution, à tort, le remboursement des créances n'est pas un, il est le remboursement d'un adieu. Finalement, toutes les entreprises sont perdantes dans cette affaire, et monsieur le ministre, j'ai bien entendu, quand vous avez expliqué il y a quelques instants que ces taxes serait exceptionnel. Mais je veux à la fois faire appel à notre mémoire et nous mettre en garde collectivement sur le caractère exceptionnel de certaines taxes en tous les cas, c'est ainsi qu'elle était promise à l'origine et qui ont connu à caractère malheureusement bien durable. à cet instant, monsieur le ministre, mais, chers collègues, je souhaiterais juxtaposées 3 chiffres étonnamment proche et qui à eux seuls, résume en quelque sorte la philosophie du gouvernement aujourd'hui un gouvernement qui pratique ce que j'appelle l'échantillonnage des 300 et quelques. 318 319, 320 318 c'est les grandes entreprises surtaxées un niveau record, 319. C'est les grandes collectivités conviés à des travaux dirigés, surveillé par l'État. Avec une forme de tutelle d'un plafond dépense et d'un ratio d'endettement mal calibré et puis 324 c'est le nombre d'emplois supprimés par l'État en 2018 sur un total de 2 millions hé bien, nous constatons avec ces 3 chiffres étonnamment proches combien les efforts demandés peuvent être variables entre les entreprises surtaxer les collectivités déjà lourdement ponctionnés par l'État et parfois à l'os et un État qui ne fait pas l'effort de se réformer en restant donneur de l'son. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous l'avez compris. Ce projet de loi de finances rectificative établi dans l'urgence, vite fait, mal fait. Nous propose de passer l'éponge sur une ardoise de 10 milliards d'euros que l'État. Avec une forme d'inconséquence. Ou d'enchaînement malheureux d'absence de décision actuellement préjudiciable aux intérêts de la France, nous propose. Eh bien, il s'agit ni plus du moins que du plus gros fiasco fiscales de l'État sous la 5ème République. Un fiasco étals d'état pardon pour lequel vous avez imaginé. En l'absence pourtant de toute responsabilité, et plus encore de toute culpabilité des entreprises, de proposer une réparation partagées à moitié. à 300 et quelques entreprises, objet d'un tirage au sort orienté. Un seul critère retenu pour être choisi, le chiffre d'affaires brut. Non corrigées de donner comme l'emploi, l'Exposition à la concurrence, la compétitivité et la profitabilité votre choix Monsieur le Ministre, est injuste. Et il augure mal aujourd'hui de l'avenir du pacte de confiance que vous appelez de vos voeux et que vous voulez par ailleurs proposé aux acteurs économiques. Nous ne pouvons le cautionner. C'est pourquoi le groupe les républicains demeurent opposés à ce projet de loi de finances rectificative et votera bien sûr la motion proposée par la commission des finances, tente à opposer la question préalable, je vous remercie. La discussion générale est Close, nous passons un discussion de la motion tendant à opposer la question préalable Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, a déposé une motion distribuée sous le numéro intendant opposer la question préalable au texte en discussion. Monsieur Albéric Dumont. Voilà bon

pour lequel le scrutin public ne m'a pas été très favorable, j'ai eu 4 voies et dès jeudi soir, donc on peut en débattre, et peut-être qu'à main levée, devant une assemblée plus nombreuses que j'ai histoire j'aurais quelques chances que cet amendement parce il est à peu dans le sens du vent non mais en tenant compte peut-être de les meilleure élasticité des recettes qui permettait de diminuer la charge d'entreprise non, plus sérieusement, je pense que le débat a eu lieu jeudi, c'est pas très clairement une position pour moi de fond qui est celle-ci s'étant largement exprimé jeudi dernier, je pense que, en le débat que nous pourrions avoir, si nous ne votons pas la commission de la la la question préalable pourrait se prolonger à l'infini, sans que les positions entre l'Assemblée nationale et le Sénat se réconcilient donc ne prolonge pas le plaisir, malheureusement, de nous retrouver, nous aurons bien sûr, nous avons du travail en commission des finances, nous avons une mission importante, celle de voter par notre collègue Gérard Longuet sur l'enseignement scolaire tout à l'heure, nous avons des missions importantes, nous sommes déjà dans le le sujet du PLF le ballon présentera pour lui mais pour sa part le PLFR demain et je pense que ces sujets nécessite un travail de fond plus importants que cette épisode donc pour moi l'essentiel aujourd'hui de tirer sur tout, comme ça a été dit à l'instant, les enseignants pour l'avenir et nous avons des enseignements trouver, c'est la raison pour laquelle je vous soumets cette question préalable, qui vise tout simplement à ne pas avoir à nouveau un débat que je considère comme largement entamé épuisés, jeudi soir, merci. Non. Contre la motion préalable, la parole est à monsieur Julien Bargeton. Je vais pas prolonger le le débat évidemment conformément à ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais voter à voter contre cette cette motion je trouve dommage moi d'écourter le débat, c'est une façon de botter en touche, peut-être que ça fait plaisir à certains de vouloir botter en touche sur ce sujet, mais je pense que ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu en terme de finances publiques et en termes de fond, si nous ne votons pas ce texte, ça veut dire que nous ne trouvons pas de solution, en réalité, ça veut dire que, il y a un ni de recettes ni de dépenses et que donc on ne répond pas à la question qui est posée, la question qui est posée, c'est que face à cette difficulté, il il faut bien trouver une solution qui soit efficace et pragmatique et donc ne pas refuser le débat et je note que, par ailleurs très souvent quand on annonce des bonnes nouvelles, ou quand il y a des recettes supplémentaires, notamment lors de notre débat sur le le projet de loi de programmation des finances publiques, on propose de l'affecter toujours et nécessairement à la baisse du difficile et à la réduction de de l'endettement, donc je pense qu'il faut être cohérent entre nos débats sur PLFR et projet de financement programmation et cela nécessite 2 donc pour maintenir le niveau, déficit public, hé bien de trouver une solution à la question qui est posée et c'est pourquoi nous nous opposons au à cette motion de rejet préalable. L'avis du gouvernement, oui, monsieur le rapporteur général. Ah dernière argument pour vous convaincre, vous savez que les intérêts moratoires court en ce moment tant à 4 04 par mois, donc si on prolongeait même que d'une heure, je sais pas quel serait le coût vu des intérêts moratoires donc

pas la vie lui armement monsieur mini-s'est exprimé tout à l'heure donc, explications de vote Monsieur Manuel qui a plus. Oui, Monsieur le Président merci juste une explication notamment sur la motivation de cette question préalable : je ne comprends pas, elle est motivée notamment pour l'par le fait qu'il que le l'Assemblée nationale aurait pas tenu compte de la position exprimée par le Sénat de quelle position parle-t-on le Sénat n'a pas exprimé position il a rejeté l'article 1 par le ton de la position des amendements Retailleau Husson et Dominati, ils ont été, qui, qui demandait la suppression de l'article 1 il a été rejeté par le ton de la position de la commission des finances et de l'amendement de monsieur de Montgolfier qui vient de le rappeler qui effectivement lui faisait une proposition

c'est que on ne peut pas sérieusement faire. L'abandon d'une discussion sur un sujet des plus sérieux, la réduction de notre déficit public et l'image de la France dans le monde et la procédure, la procédure c'est une 2ème raison qui fait que on ne peut pas faire l'économie du débat, même si je suis d'accord avec le rapporteur, j'aime général on a fini un peu tard jeudi soir et la 3ème raison c'est que on ne peut pas non plus motivé une question préalable par le fait de dire que on a peu d'espoir de faire revenir l'Assemblée nationale a des positions qui sont plus conformes à la nôtre parce que dans ces cas-là, il faut fermer la boutique et nous n'avons plus de raison d'être, donc pour l'ensemble de ces 3 raisons, et à l'unanimité, le groupe des Indépendants votera contre la question préalable. y a, il y a pas d'autre explication de vote, je vais mettre aux voix la motion numéro 1 de monsieur Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, on aura opposer la question préalable, je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi de finances rectificative pour 2017 je rappelle en août que l'avis du gouvernement, exprimé dès la les explications et et défavorable en application de l'article 51 du règlement, le scrutin public ordinaire et de droit, donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin va être ouvert dans quelques instants.

Le scrutin est ouvert.

le scrutin est clos invité secrétaire du Sénat à procéder au dépouillement du scrutin.

Résultat du scrutin sur la motion numéro 1 tendant à opposer la question préalable contenu l'ensemble de délégations de vote accordé par les sénateurs, politique et notifié à la présidence. Nombre de votants : 342 Nombre de suffrages exprimés 341. Pour l'adoption 146 contre 195, le Sénat n'a pas adopté. nous passons à la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2017. Sur la première partie conditions générales de l'équilibre financier, je vais mettre, on voit donc l'article 1. Monsieur Guillaume pour explication de vote. Le président, monsieur le ministre est-ce que vous nous accorderez de suspension de séance.

Donc, la séance s'est reprise. Donc je de nouveau. On voit l'article à Monsieur Reina l'explication de vote. Oui, Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, simplement par rapport à ce que j'ai avancé tout à l'heure, je voudrais peut-être mieux préciser les choses, il me semble qu'il y a 2 questions qui nous sont posées : une première qui ne nous convient pas, nous le rappelons mais qui aujourd'hui a été voté par notre assemblée qui est l'article 5 sur le décret d'avance : nous avons combattu tous les éléments de ce décret d'avance et donc ce décret d'avance a été approuvée par notre assemblée nous le, nous le regrettons concernant ici la question de la taxe je voudrais pas et nous ne voudrions pas qu'il y a de confusion, car effectivement on voudrait pas que, il y a une confusion entre la position, NDLR d'opposition à cette taxation et notre position qui est simplement de dire que nous regrettons que dans le cadre cadre actuel qui nous est proposé un certain nombre d'entreprises qui n'étaient pas touchés, en particulier l'entreprise mutualiste le soir le soit aujourd'hui notamment, c'est un point qui nous paraît extrêmement important de ne pas avoir non plus une vision complète des gagnants et des parlant, pour faire simple, dans la formulation nous paraît une faiblesse, mais en même temps nous n'ouvrirons pas mêler nos voix mêlées des voies d'abstention et des voix d'opposition donc ce que nous vous proposons ce que nous vous disons, c'est que le groupe socialiste votera l'article par contre du vote qui a été fait sur l'article 5 en tout cas sur l'article qui nous est proposé, nous voterons pour aller dans le sens de la, de l'intérêt de notre pays, nous voterons l'article 1.

de vote. Monsieur Salvador oui. Merci monsieur le président, chers collègues, comme on a un esprit de suite et une cohérence, vous comprendrez que nous ne participeront pas au vote sur l'article 1, 1, nous voterons contre l'article 5, particulièrement pour les mêmes raisons que le sénateur et mal à l'expliquer et que ça marche pas le micro. Ah non, mais c'était j'écoute et que nous voterons contre le texte in fine. Monsieur Dominati. souvent pour quelques instants, le débat sur le fond, je rappellerai simplement très rapidement les 3 raisons qui ont amené le groupe républicain voter contre ce texte, tout d'abord sur le fond, cette taxe sur les dividendes, c'est une mesure faite par le président Hollande une mesure socialiste une mesure emblématique et ça explique probablement le revirement du groupe socialiste sur cet article 1 puisque c'était la mesure emblématique disant mon ennemi c'est la finance donc le réflexe immédiat avait été de taxer les entreprises et les entreprises les plus performantes ou les plus grandes du pays 2ème argument: c'était la stabilité fiscale, le nouveau président de la République, le nouveau gouvernement disait les choses ont changé, on a compris que ce pays avait besoin et le monde économique de stabilité fiscale et moyennement en quoi en 5 semaines, au moment où toutes les entreprises ont prévu leur budget, leur politique vis-à-vis de leurs actionnaires, ne trouvant pas d'autres chiffres dans l'urgence ont décidé de faire sur cette stabilité fiscale et tout ce qui, dans cet hémicycle à longueur de débats réclame la stabilité fiscale embrayé en 5 semaines en disant 5 milliards, on les trouve comme ça, c'est pas grave c'est les grandes entreprises et le monde de l'entreprise qui va payer au-delà la stabilité fiscale, on dit il y a pas d'autres mesures proposées un certain nombre d'autres mesures ont été proposées au moment où le gouvernement parle de privatisation, on parle de Prévit Aviation fait par des entreprises publiques, il y aurait peut-être une solution, monsieur le ministre vous l'a proposé et lorsqu'on dit, l'Assemblée nationale n'a pas tenu compte du débat du Sénat, c'est vrai, il pouvait peut-être y avoir de la part du gouvernement, d'autres propositions, enfin, au moment où il y a eu le Brexit, où la place financière de Londres est concurrencé maintenant par la place financière de Paris et celle de Francfort, au moment où un certain nombre d'autorité, comme le 1er ministre, le président de la République, on parlait de mesures nouvelles, cette mesure va totalement à contre-sens, on dit c'est une exception et cette exception elle n'a même pas compenser au cours de l'exercice prochain si le gouvernement nous avait dit il y a une urgence et pendant quelques semaines facialement même si soi-disant surnom la sincérité, on va essayer de tenir les coûts vis-à-vis de Bruxelles, et bien on compensera l'an prochain, vis-à-vis du monde de l'économie et vis-à-vis du des entreprises, ce n'est absolument pas le cas, ces mesures d'exception, effectivement, il y a une philosophie il y a une éthique et synthétique ici n'est pas respecté, c'est automatiquement le monde de l'entreprise et le monde économique qui est la vache à lait, dès qu'il y a un souci dans les finances publiques et une imprévision dans les finances publiques, donc c'est une faute gouvernementale qui a été faite par le président lors des vient 5 ans et c'est une double faute qui est faite aujourd'hui par ce nouveau gouvernement. Pas d'autres explications de vote, donc je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains ont il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est clos.

Donc, voici les résultats du du scrutin quand tu l'ensemble délégation de vote accordé par les sénateurs ou politique et notifié la présidence. Nombre de votants : 325 Nombre de suffrages exprimés 315 pour l'adoption 171 contre 144 donc, l'article 1er est adopté. Je mets au bois, l'article 3. Donc, l'article 3 qui est favorable, c'est là une des conséquences de l'article 1er, monsieur le rapporteur. à l'accord, pardon, donc là, l'article 3 qui est favorable, article 3.

Oui, d'accord, les autres dispositions de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2017 ne font pas l'objet de la nouvelle lecture, je vais mettre aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2017, je rappelle qu'en application de l'article 40 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de l'article 47 bis alinéa 2 du règlement lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finance l'ensemble du projet est considéré comme rejeté, y a-t-il de demandes d'explications de vote. La demande d'explication de vote. Je mets au voix l'ensemble de la première partie du projet de loi. Qui est favorable.

Donc la première partie du projet de loi est adopté. Les autres dispositions de la 2ème partie du projet de loi de finances rectificative pour 2017 ne font pas l'objet de la nouvelle lecture. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Appartient et 2ème partie. je je mets, on voit le le projet de loi de finances rectificative pour 2017. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public et de droit, donc il va être procédé dans les conditions fixées par article 56 du règlement. Le

Le scrutin est ouvert.

Donc, voici les résultats du scrutin, donc sur l'ensemble du texte, compte tenu des délégations de vote accordé par les sénateurs groupes politique et notifié la présidence Nombre de votants : 342. Suffrages exprimés 263 pour l'adoption 102 contre 161 donc, le Sénat n'a pas adopté. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux afin de s'il vous plaît. Juste une seconde, une seconde attention avant la suspension de séance, nous allons interrompre nos travaux afin de permettre la tenue de la cérémonie d'hommage à Georges Clémenceau dans le salon des messagers d'État à séance reprendra à l'issue de cette cérémonie à 16 heures 40 pour poursuivre poursuivre cet hommage en séance publique, puis les questions d'actualité au gouvernement, la séance est suspendue.

Monsieur le 1er ministre. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Il y a un siècle. Le 16 novembre 1917. Georges Clémenceau, sénateur du Var, président de la commission de l'armée au Sénat, a été nommé président du conseil par le président Raymond Poincaré. Poincaré. Paraît alors à bout de force. Les morts. Se comptent par centaines de milliers. Les combattants sont épuisés. Des mutineries éclate. L'arrière est affecté par des grèves et des pénuries alimentaires. Alors que le doute s'installe, Georges Clémenceau rassemble toutes les énergies du pays en vue de la victoire. Combatifs, déterminés, il résume son objectif sur le plan intérieur comme extérieur en un seul mot, un seul mot d'or, je fais la guerre. Le président du Conseil, accompagné de son chef de cabinet, Georges Mandel multiplie les visites dans les tranchées, ignorant les balles qui sifflent autour de lui. Sous le regard d'abord étonné puis admiratif des soldats déployés. Georges Clémenceau restaure alors la confiance et de courage, non seulement des troupes, mais aussi des élites politiques et intelectuelles tentés par le défaitisme, dès lors, ce travailleur infatigable consacre chez jours et ses nuits à son combat, il il ne quitte son bureau de la rue Saint-Dominique, que pour le front et pour le Parlement, accompagné de son sous-secrétaire d'État à la guerre, Jules Jeanneney, qui deviendra par la suite, président du Sénat en 1932 il soumet ses actes au contrôle des commissions des 2 assemblées, il ne fut jamais les débats publics et affronte la question de confiance qui lui est à chaque fois accordé, il répète qu'il n'a de compte à rendre qu'au président de la République et aux chambres. Le 17 septembre 1918 dans notre hémicycle ici même, il déclare : que voulons-nous combattre combattre victorieusement encore et toujours, jusqu'à l'heure où l'ennemi comprendra qu'il n'y a plus de transactions possibles entre le Crime et le droit. Maréchal Foch lance alors 3 offensives qui seront déterminantes. Le 11 novembre 18, cet homme de 77 ans, courbé monte à la tribune de l'Assemblée pour annoncer la victoire grâce à lui, la France retrouve sa place dans le monde pour poursuivent, dit-il alors sa course magnifique pour le progrès humain. Il allume cette place de la Résistance, cette flamme de la Résistance qui ne s'éteindra pas. Le 11 novembre 1941 de Londres le général De Gaulle s'adresse à Georges Clémenceau et je le cite. Au fond de votre tombe vendéenne Clémenceau vous ne dormez pas car la vieille terre de France qui vous en terre pour toujours tressaillir avec colère tandis que le Lepage selon de l'ennemi et la marche feutré des traites foulé le sol de la patrie. Quand la victoire sera gagnée et que justice sera faite, les Français viendront vous le dire, alors avec tous les morts dont est pétri la terre de France vous pourrez dormir en paix. Charles de Gaulle le 12 mai 1946 il y a, se recueillir sur sa tombe à mouchant en Vendée et il y a en quelque sorte lui annoncer la victoire. C'est une fois encore, la victoire du courage face au renoncement ce courage dans nos soldats font preuve aujourd'hui au Sahel au le et au quotidien sur le trottoir de France, de ces jeunes tombés dans les sables du désert tout comme leurs frères d'armes du même âge, tombé il y a un siècle en Artois dans la Somme à Verdun, il ce courage, nous le devons à Clémenceau qui su faire vibrer au sein de notre hémicycle ce véritable élan non. Je reprends sa forme, il n'y a plus de transactions possibles entre le Crime et le droit. C'était vrai hier c'est vrai aujourd'hui, voilà le message de Clémenceau.

Merci, mes chers collègues. Reprises. Monsieur le 1er Ministre Mesdames et messieurs les ministres, cher collègue, l'envoi du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement, la séance est retransmise en Direct sur Public Sénat sur notre site Internet et sur Facebook chacun portera les valeurs essentielles du Sénat dans ces temps de débats et d'échanges, le respect des uns et des autres et d'une manière pragmatique, le respect du temps, la parole est maintenant notre collègue Madame Esther ben ça pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Thierry Carcenac est disponible pour le groupe socialiste et républicain, je remercie, je l'invite à poser sa question. merci monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'action et des Comptes publics, monsieur le ministre vous avez confirmé l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source, levant ainsi une incertitude sur l'avenir de la réforme engagée par le précédent gouvernement, c'est une excellente nouvelle qui constitue une modernisation sans précédent du recouvrement de l'impôt sur le revenu pour nos concitoyens, elle permet de rendre le paiement de l'impôt, contemporain de la perception des revenus, c'est également une mesure de justice qui protège ceux dont le revenu évolue chaque année 30 pourcent des des contribuables sont concernés, toutefois, monsieur le ministre, suite à votre annonce ce lundi à Toulouse, il demeure quelques interrogations : la mise en place au 1er janvier 2019 ça inscrira-t-elle dans la continuité du dispositif prévu par le précédent gouvernement dans les objectifs était, je le rappelle, l'adaptation de l'impôt, la vie professionnelle de nos concitoyens, ainsi qu'une meilleure répartition de l'impôt dans leur nez puisqu'elle sera désormais étalé sur 12 mois, autre interrogation suite à votre annonce le coût pour les entreprises, en effet, vous aviez justifier le report d'un an de la mise en place du prélèvement en raison d'un coût insupportable pour les entreprises, j'espère qu'aujourd'hui, ce problème est résolu, sachant que dans le dispositif initial, il était prévu le déploiement de la déclaration sociale nominative dont on nous dit aujourd'hui que sa mise en oeuvre se passe dans les meilleures conditions, autre interrogation : pouvez-vous confirmer la division par 2 de l'amende applicable en cas d'erreur de la part des employeurs, telle que vous l'avez indiqué lundi cette annonce sera en effet de nature à rassurer les entreprises et plus particulièrement les plus petites, enfin, qu'en sera-t-il de l'armée blanche cette disposition concerne a raté l'ensemble des revenus, ce qui aurait le mérite de la simplicité, où allez-vous prévoir des dispositifs dérogatoires qui entraîneront complexité et donc sur ce dernier je vous remercie. De l'action et des Comptes publics monsieur Gérald Darmanin vous avez la parole Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur le sénateur, comme vous l'avez évoqué et suite débat que nous avons ici au début de la nomination du gouvernement, nous avons donc confirmer effectivement qu'au 1er janvier 2019 après un an de de report l'impôt à la source, sera mis en place et je voudrais ici remercier tous les agents de la DGSI qui ont travaillé sous l'ancien gouvernement comme celui-ci pour que cet impôt qui est recouvert, aujourd'hui l'impôt sur le revenu par 98 98 pourcent puisse puisse se faire dans les meilleures conditions de simplicité effectivement au service des contribuables dont quasiment la moitié de ceux qui payent l'impôt sur le revenu voir leurs revenus fluctuer et je pense que c'est une mesure de de simplicité pour cependant, nous avons eu raison monsieur le sénateur, on a eu ce débat, rappelez-vous de reporter d'un an à la demande du 1er ministre la mise en place de cet impôt la sur ce rapport de l'Inspection générale des finances et du cabinet Mazars prévoit en effet que si nous avions mis en place au 1er janvier 2018 l'impôt à la source, rue de graves risques de défaillance et je crois que c'était pas à mettre du côté des agents de la fonction publique mais bien devant la révolution que vous évoquez de simplification de de cet impôt 2ème sujet : nous avons fait une phase de tests en en grandeur réelle avec plus de 600 entreprises à Toulouse, je suis allé avec beaucoup de vos collègues, rencontrer une des entreprises qui avaient quelques centaines de de salariés qui a mis en place, face de 600 collecteurs, les collectivités locales, les associations employeurs, les entreprises et cette phase test à des conclusions qui nous permettent quand même d'améliorer ce dispositif alors il y avait un rapport sénatorial qui, plus d'un 1000000000 de coût pour les entreprises,

hé oui, nous allons prendre des mesures dans le débat parlementaire et je serai très ouvert aux amendements pour simplifier la vie des entreprises, notamment des petites d'entre elles afin de réduire le plus possible ce et rendent ce service à nos concitoyens. 9 secondes. Mots pour partager avec monsieur le ministre, le remerciement du grand professionnalisme des agents des impôts. Merci, la parole est maintenant à notre collègue Esther Ben Basat pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologique avait la parole, ma chère collègue. Merci monsieur le président, Monsieur le Président mais chers collègues bien et les autorités israéliennes ont annoncé qu'elles refuseraient l'entrée sur leur territoire territoire d'élus français, dont 7 parlementaires issus des diverses gauche qui s'apprêtaient auront à se rendre à l'Israël pour porter un message de paix et de femmes, actualité et afin d'alerter sur la situation des prisonniers politiques palestiniens,

d'entrée serait d'abord le soupçon supposé soutien de la délégation au mouvement international boycott, désinvestissement sanctions connu sous le nom de B. qui vise à dénoncer et à punir la poursuite de de l'occupation en Cisjordanie le soutien supposé des responsables politiques concernés au PDS est loin de constituer une menace pour Israël et il relève des convictions personnelles de chacun, il s'agit de prétexte de dernière minute, vu que ce voyage initiée par l'Association Jumelage Palestine France AJPF avait été préparée en collaboration avec le consulat français de Jérusalem : que compte faire le gouvernement français pour remédier à cette décision inique. Pour vous répond : la parole est. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoine, c'est le ministère de la parole. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame Massin tristesse termine ça effectivement, comme vous l'indiquez, les autorités israéliennes viennent d'annoncer qu'elle n'autoriserait pas des parlementaires français parlementaires européens à venir dans le cas de la visite organisée par une association, association qui avait annoncé qu'elle se rendrait avec un certain nombre de ses parlementaires pour rencontrer Marwan Barghouti et Salah Hamouri tous 2 emprisonnés alors on peut regretter cette décision israélienne, elle en reste néanmoins souveraines alors de façon générale, nous souhaitons la France souhaite ardemment que les parlementaires puissent avoir accès aux personnes qu'souhaitent rencontrer lors de l'année, lors de leurs déplacements, que ce soit à et Israël ou dans les autres pays du monde naturellement notre consulat général d'ailleurs était intervenu pour appuyer cette demande de la même façon que notre consulat général et mobilisée au quotidien, je peux vous le dire, s'agissant de la situation de Salah Hamouri, il lui a rendu visite sur son lieu de détention, il a assisté à l'ensemble des audiences publiques auxquelles il a comparu et nous avons signalé aux autorités israéliennes, je peux vous le dire, pour l'avoir fait personnellement toute l'attention que nous portons à ce cas parce que il pose un problème plus large qui est le recours extensif à la détention administrative, ce qui fait que nous ne savons pas, d'ailleurs, quels sont les griefs qui sont retenus contre Monsieur Salah Hamouri, instamment aux autorités, hé bien, le respect de ses droits, naturellement, nous espérons que sa libération puisse intervenir et donc vous le voyez madame la sénatrice, nous sommes pleinement mobilisés et j'ajouterai que cela ne doit pas nous décourager et que la France continue à porter aussi une parole de paix d'apaisement avec d'initiatives culturelles, que ce soit dans les territoires palestiniens, ouverture d'un lycée français à Ramallah ou bien avec la saison culturelle croisée France-Israël et nous espérons que ce seront des ferments de paix et de compréhension, je vous remercie. Alain Massa pour 15 secondes. En refusant l'entrée de cette délégation à l'Israël, le gouvernement de Binyamin Nétanyahou ne fait que confirmer que les efforts pour la paix Nantes pas actuellement dans ses objectifs : la France me semble-t-il, ne devrait pas devenir complices en optant pour le silence. Merci, la parole est maintenant à notre collègue Jean-Louis Lagourgue pour le groupe, les indépendants républiques et territoires, vous avez la parole, mon cher collègue, pour 2 minutes. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la transition écologique et solidaire. Monsieur le Ministre, vous le savez, la ville de Bonn accueille actuellement la pop 23. Dernière échéance en date des négociations internationales sur le changement climatique. Indolent le collègue du groupe Jérôme Bignon, il y a d'ailleurs actuellement pour participer au débat. C'est un rendez-vous international de première importance, Bill puisqu'il vise à définir les modalités pratiques d'application de l'accord climatique de Paris signé à l'issue de la COP 21, malheureusement, l'engagement de limiter le réchauffement global est aujourd'hui menacé menacé d'abord par la décision de l'administration américaine de se retirer de cet accord au risque de fragiliser le consensus international sur leur agence climatique menace ensuite par la difficulté technique à tenir le franc engagement d'un réchauffement climatique limiter à 2 degrés à l'horizon 2100 le 30 octobre dernier à l'occasion de son rapport annuel sur les perspectives de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'ONU a présenté une simulation n'réchauffement autour de 3 degrés, cette situation a des conséquences directes pour notre environnement conséquence exposé lors de l'examen du projet de loi sur les hydrocarbures, nous avons ainsi invoquer ce qu'une hausse du niveau des mers signifierait pour notre pays, transformation de la Camargue de l'estuaire de la Gironde et autres, et bien entendu engloutissement des codes d'une large partie de nos territoires ultramarins dans le département de la Réunion, il faut donc agir vite et il ne faut pas baisser les bras tout au contraire, il faut redoubler d'efforts pour promouvoir des énergies propres et des pratiques, durables, le territoire de la réunion a été ainsi pleinement engagé dans cet effort de transition énergétique de de la production électrique locale et fondée sur les énergies renouvelables, les droits, il faut conclure, c'est pourquoi monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser les mesures que vous entendrez pour poursuivre la transition énergétique et ne pas manquer le virage de cette révolution des mentalités et des pratiques. Pourrait prendre la parole est au secrétaire d'État. Près du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire monsieur le nu, monsieur le ministre avait la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, permettez-moi d'excuser le ministre d'État, Nicolas Hulot qui se trouve effectivement actuellement à la COB 23 où il porte la voix de la France, vous avez raison Monsieur sénateur, il y a urgence à agir en matière de transition écologique en matière de transition énergétique, c'est ce que les scientifiques hier ont rappelé dans le journal Le Monde, mais la France d'outre-mer, n'a pas besoin qu'on lui rappelle puisqu'elle vit très directement les dérèglements climatiques, vous le savez vous-même à la Réunion, le 1er ministre était dernièrement avec une délégation de 6 ministres, aux Antilles et nous avons encore pu constater à quel point l'avancée du trait de côte, le montée du niveau de la mer est un sujet extraordinairement préoccupant : la réponse de la France et du gouvernement depuis le mois de mai dernier, agit sur 3 volets d'abord évidemment le volet international, c'est la participation de la France à la com 23 c'est le Pacte mondial pour l'environnement en septembre dernier à l'Assemblée générale des Nations unies s'est également bien évidemment le sommet du 12 décembre prochain pour fêter en quelque sorte l'anniversaire de l'accord de Paris mais le rendre opérationnel et parler très clairement des financements à l'heure où les États-Unis d'Amérique se retire peu à peu de cet accord, il y a aussi bien évidemment à voler national le plan climat Nicolas Hulot qui l'a proposé et présenté aux Français au mois de juillet dernier, le projet de loi portant interdiction de l'exploration et l'exploitation hydrocarbures que vous avez discuté récemment les mesures de transition pour les Français, y compris des Français les plus modestes pour leur logement ou pour leur voiture, la préparation d'une prochaine programmation pluriannuelle pour l'énergie, avec un nouveau mix énergétique, pour lequel le gouvernement souhaite que le Sénat soit étroitement dans sa préparation, bref la réponse nationale est ambitieuse et vous l'avez dit, monsieur le sénateur, il y a une réponse, c'est pour cela que le 1er ministre a validé une enveloppe exceptionnelle de 75 millions d'euros pour répondre à l'urgence pour les territoires énergie positive pour la croissance verte pour lequel il y avait une difficulté de financement, c'est pour cela que nous développons les contrats de transition écologique pour l'année prochaine, la réunion d'ailleurs pourra y candidater monsieur le sénateur, et c'est pour cela que nous souhaitons développer les énergies renouvelables, en particulier dans les outre-mer, c'est le souhait également de Madame Girardin, merci à tous. Merci monsieur le ministre, la parole est à notre collègue.

chaque vendredi dans Les Hauts-de-Seine à Clichy chez d'autres collègues, Rémi Muzeau que plusieurs centaines de musulmans envahissent le trottoir pour faire leur prière, juste en face de la mairie qui est tout de même le symbole de la République, cela fait 8 mois que ces personnes refusent d'occuper des lieux qui pourtant sont prévus à cet effet, sous des prétextes les plus fallacieux qui soit et cela fait 8 mois que l'État ne fait rien et laisse ce territoire abandonné et il a fallu que une centaine d'élus se manifeste et au Champ de la Marseillaise fasse reculer cette abandon du du territoire alors Monsieur le ministre ma question est simple est-ce que vous comptez oui ou non faire quelque chose pour faire cesser cette situation et est-ce que vous comptez faire en sorte que les élus demain n'aient plus à se substituer aux forces de l'ordre pour tout simplement faire respecter l'ordre républicain, merci Monsieur le midi. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur avait la parole, Madame la Ministre. Merci monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, c'est. Vous avez rappelé ce qui se passe effectivement à Clichy, à la suite d'une décision de justice, l'une des 2 salles de prière que comptait la ville de Clichy a été fermée le 22 mars dernier depuis des prières de rue sont organisés par l'ancienne association gestionnaire d'abord sur un rythme quand il y a un désormais sur un rythme hebdomadaire, personne ne peut se satisfaire de cette situation. Il revient au ministre de l'Intérieur de rêve de veiller au respect de la loi. Au sens général à Clichy, il y a une décision de justice qui autorise la mairie a affecté les locaux de la rue d'Estienne d'Orves à d'autres finalités cette décision de justice doit être respecté, le week-end dernier, le maire de Clichy-la-Garenne, a fait part de ce qu'il y avait eu des prêches avec des appels aux meurtres et des tracts antisémites diffusés à l'occasion des prières, monsieur le sénateur, ce n'est pas une provocation, ce que je vous dis mais fait l'État n'a pas connaissance de ces documents, j'invite donc tous ceux qui disposent de telles informations. En faire part à la justice et au service de l'État, auquel j'ai demandé de maintenir la plus grande vigilance dans le respect des conditions fixées par la loi de 1905, il faut bien sûr que toutes les religions puissent exercer de façon constante convenable leur culte, une piste possible pour trouver un nouveau local pour l'association vient malheureusement d'échouer, il y a quelques jours, j'ai demandé aux préfets de poursuivre son travail en ce sens pour mettre très rapidement un terme définitif à la situation actuelle, mais monsieur le sénateur, pour mettre fin à Toulouse cette situation nous comptons aussi bien sûr sur le maire de Clichy, car le maire de Clichy et le ministre de l'Intérieur doivent travailler de concert pour trouver une solution à se suivent problème. croyais madame je croyais, Madame la Ministre, que nombre d'élus était une utile mais je vois qu'en permanence vous faites appel à vous n'avez pas les mêmes informations, je vous rappelle qu'à Clichy, il y a une église, une, 2 églises et synagogues et de lieux de prière pour les musulmans, je crois que nous avons tout simplement pas la même conception de l'ordre public et pourtant un certain nombre de ceux qui sont ici ont été maire avant d'être ministre, la réalité, vous la connaissez, à certains endroits, en fait, on nous sommes envahis par le fait religieux, et cela provoque nos convictions, quelle qu'elle soit, cela provoque la liberté et notre démocratie, alors Madame le Ministre, Mesdames et messieurs du gouvernement, j'en appelle à vous pour restaurer la République en tous lieux, des territoires, parce que, selon moi, la République est selon vous aussi j'imagine la République elle est une et indivisible. Merci. La parole est maintenant notre Collègue Olivier et nous pour le groupe de l'Union centriste, vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le président, Monsieur le 1er Ministre Mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires depuis plusieurs mois, nous attendions de la part du président de la République et du gouvernement une vision et des perspectives en matière de politique de la ville, en effet, il est toujours plus pertinent avant de démolir ou de passer un coup de rabot financier de préciser sa vision de définir une alternative et surtout d'organiser un débat national pour que cette alternative, soit la plus féconde possible, le président de la République, en déplacement dans le Nord, a fait quelques annonces sur ce que nous pouvons considérer comme un énième plan en faveur des quartiers et territoires cumulant de nombreuses difficultés urbaines, sociales, de sécurité et l'emploi, certaines pistes annoncées semblent sortis de ce que certains appellent l'ancien monde ce qui pense ça, d'ailleurs, je les invite à lire ou relire les clés Zia comment comprendre la création d'emplois francs quant au même moment les collectivités et les associations des mêmes quartiers doivent faire face à des disparitions de contrats aidés, des annonces ont été faites en matière d'éducation de culture de lutte conte la discrimination et d'accès aux services publics, nous les partageons ces annonces attendue par de nombreux acteurs dans nos territoires, laisse quand même un goût de trop peu alors quelle vision en matière de sécurité, de logement et de service public de l'emploi, et enfin quelle place et quel concertation avec les territoires et leurs élus locaux, il n'y a pas de fatalisme dans le domaine de la politique de la ville et j'encore à l'esprit les 2 Métamorphose des quartiers qui avait suivi le plan de Jean-Louis Borloo, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, éclairez notre assemblée sur la vision à court, moyen et long terme en faveur des quartiers des territoires les plus fragiles de notre République.

président de la République s'est expliqué très clairement sur sa vision de la politique de la ville qui est celle de tout le gouvernement et il l'a fait en concertation avec bien sûr le 1er ministre et l'ensemble du gouvernement, c'est un enjeu considérable, un enjeu considérable et ce qui se passe dans nombre de quartiers n'est pas le résultat de la politique qui est menée depuis 5 mois, c'est ce qui c'est le résultat de 50 de ce au moins 50 années au cours desquelles malheureusement un certain nombre de quartiers ont été marginalisés avec aujourd'hui des constatations qui sont malheureusement difficiles. Avec des problèmes de sécurité avec des problèmes d'emploi, avec des problèmes d'éducation vous avez cité, Jean-Louis Borloo, nous avons pris, nous mais, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Ministre, vous qui connaissez bien aussi l'cette politique-là, nous avons décidé de confier une mission à Jean-Louis Borloo, qui va travailler avec moi et avec le secrétaire d'État, Julien, de Normandie, nous avons voulu et c'est l'expression du président de la République, avoir une vision de rassemblement dans un dossier qui est une priorité nationale au nom de ce rassemblement, nous avons pris aussi la décision de nommer Monsieur Klein, maire socialiste de Clichy, président de l'ANRU car il est nécessaire dans ce débat extrêmement important de rassembler le Max toutes les sensibilités, car il y a là une véritable priorité nationale, vous avez rappelé tout à l'heure, ce qui se passe dans certaines communes avec le retrait de la République avec des comportements que nous ne pouvons tolérer ou que nous soyons assis sur ces bancs, quelles que soient nos sensibilités, et c'est le message très fort qui a diffusé, le président de la République en indiquant d'ailleurs que tous les 3 mois, il veillerait à réunir autour de lui à l'Élysée, dans une réunion de travail, les acteurs de la politique de la ville pour faire le point, pour avancer en totale bien sûr concertation avec le 1er ministre et l'ensemble du gouvernement, c'est une vraie politique de relance de la politique de la de la ville telle qu'elle n'avait pas été envisagé depuis bien longtemps. Monsieur le président, Mesdames et messieurs, le les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mahdia Madame Agnès Buzyn, ministre des solidarités, de la santé et cancer ne les dispositions du PLFSS concernant la prévention des cancers de l'utérus, fait, c'est ce que nous étudions en ce moment même au Sénat, prévoit de nombreuses innovations je tenais Madame la ministre a salué la position du gouvernement pour agir en faveur d'une meilleure prévention des cancers. Selon les recommandations de la chasse, le dépistage commence chez les femmes à 25 ans pour le cancer du col et à 50 ans pour celui du sein et du colon, dans le cadre de la prévention des cancers féminins, la mise en place d'une consultation spécifique et sa prise en charge à 100 pourcent par par la Sécurité sociale pour les assurés âgés de 25 ans est essentielle pour diffuser les messages de prévention et permettre un dépistage effectif de la population, cette consultation offrira en plus d'un dépistage du cancer du col de l'utérus à l'ensemble de la population d'identifier dans la population féminine, les patientes qui aurait besoin d'un dépistage plus précoce avant 50 ans pour le cancer du sein par exemple si je salue donc votre initiative, l'âge de 25 ans pourrait paraître trop tardif pour Dave en prévention primaire, en effet, les outils à disposition de tels que le vaccin anti-papillomavirus du col de l'utérus en démontré leur efficacité, car à administré à des jeunes filles plus jeunes 12 ans dans une récente étude au Royaume-Uni pour cette raison, je souhaiterais connaître madame la Ministre votre sentiment sur l'instauration d'une première consultation de prévention pour les assurés entre l'âge de 11 et 14 ans pour faciliter la discussion autour du vaccin, mais pas seulement, et rappelle éventuellement l'utilité de l'activité physique du contrôle de la charge pondérale et l'évitement de la toxicomanie. Non, répondent la parole, ça va dames la ministre. Des solidarités, de la santé Madame Agnès Buzyn, vous avez la parole. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous avez raison, la prévention doit être une doit être une priorité et nous avons instauré dans le PLFSS une consultation de creux 11 une consultation de prévention gratuite pour les femmes âgées de 25 ans afin d'identifier leur niveau de risque pour les cancers du sein, de façon à ce qu'elles bénéficient d'un dépistage plus précoce et afin de les alerter sur l'utilité du dépistage du cancer du col de l'utérus par frottis puisqu'aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus seraient totalement évitables si l'ensemble des femmes françaises se soumettent à un frottis tous les 3 ans. Par ailleurs, il existe une prévention primaire par la vaccination anti-appelle HPV et de nombreux pays, notamment l'Angleterre, l'Australie, on fait des grandes campagnes de vaccination chez l'ensemble des enfants, fille ou garçon, depuis 2007, ce qui a permis une diminution de la prévalence du virus et une diminution de la prévalence du cancer du col et des lésions du col utérin chez 75 pourcent des des femmes en Australie, ce qui a été vraiment prouvé scientifiquement comme une excellente mesure de prévention primaire, la question qui se pose donc à notre pays est une large campagne de vaccination contre le virus HPV pour les filles comme pour les garçons, cela permettrait d'une part de faire diminuer la prévalence du virus atypique à ce PV dans la population et, d'autre part de prévenir chez les jeunes garçons d'homosexuel, le cancer du Canada, ainsi que les cancers ORL, il faut donc avoir une réflexion plus générale sur la consultation de prévention que l'ombre, mettre en place pour favoriser la vaccination de l'ensemble de nos jeunes pour le virus HPV, par ailleurs, vous avez raison, nous devons nous interroger sur l'intérêt d'une d'un dépistage de précoce de l'obésité, c'est la raison pour laquelle, avec Jean-Michel flanker nous voulons rendre effective la visite médicale à 6 ans pour tous les enfants de façon à dépister notamment le surpoids et l'obésité, donc nous avons une réflexion très large sur l'ensemble des consultations de prévention nécessaire pour être utile aux Français, et nous avons ouvert ce débat aujourd'hui sur la vaccination HPV, mais de façon plus large que simplement la vaccination des jeunes filles, je vous remercie. La parole est à notre collègue Joël Labbé pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, si ministre, pardon mesdames et messieurs les Ministres, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, chers collègues, d'abord, je suis très très déçu que le ministre de l'agriculture ne puisse être là, j'aimerais bien poser mon joker, mais ça ne se fait pas, alors je je voudrais interpeller le gouvernement concernant le soutien à l'agriculture biologique. En ces temps où l'agriculture dite conventionnelle démontre ses limites au point de ne plus nourrir ses serviteurs, que sont les agricultrices et les agriculteurs une un nombre de plus en plus grande de paysannes et paysans choisissent d'engager une transition vers l'agriculture biologique mieux rémunératrice pour les producteurs plus vertueuses, tant pour la fourniture de productions de qualité, de préservation de la vie des sols déséquilibres environnementaux de la biodiversité de la qualité des eaux de la santé humaine, du climat et j'en passe

des des aides de la PAC, qui se chiffre, je vous le rappelle, à 7,44 milliards d'euros annuels alors et vous, enfin vous lui direz Monsieur le Ministre de l'Agriculture, vous avez décidé, pris la décision que l'État se désengage des aides au maintien pour se recentrer sur les aides à la conversion estimant je estimant que, je le cite le ministre de l'Agriculture, c'est désormais au marché de soutenir le au au marché de soutenir le marché de l'agriculture biologique, votre message, monsieur le ministre est absolument inacceptable et incompréhensible, cela alors que le président de la République a annoncé la reconnaissance de la valorisation des services environnementaux, produit par les agriculteurs à travers un avertissement de 200 millions d'euros pour mettre en place rapidement des paiements pour services éco-systémiques alors ma question, monsieur le Ministre ou Madame la Ministre, qui va, qui va vous qui va pouvoir me répondent, qu'en est-il de ce financement annoncé par le président de la République

Monsieur. Le corps du secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique va vous répondre. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur la je vous rassure le ministre à travers une bonne raison de ne pas avec nous cet après-midi pour cette séance de questions gouvernement puisqu'il est, avec l'ensemble des acteurs d'une filière pour justement négocier une juste répartition de la valeur entre transformateurs et distributeurs, donc je vais donc fidèlement vous apporter sa réponse est sous l'autorité du 1er ministre celle du gouvernement, je vous confirme que l'action du gouvernement vise à conforter accompagné monsieur sénateur la filière bio, vous le savez, nous avons fait le choix en juillet dernier d'un transfert de crédits du pilier de la politique agricole commune vers le pilier 2 pour poursuivre poursuivre et zou du nos actions en faveur du bio et des agriculteurs les plus fragiles, car nous sommes trouvés devant une impasse budgétaire et nous avons souhaité que les aides au bio ne soit pas la variable d'ajustement par ce transfert nous garantissons les aides à la conversion dans la dynamique de croissance qu'elles connaissent, nous confions désormais aux conseils régionaux le soin de continuer à financer des aides au maintien sur nouveau contrat mais elles devront le faire en responsabilité et sans mobiliser les crédits de l'État, outre ces aides à la conversion, les agriculteurs bio bénéficient de mesures agro-environnementales, il bénéficie naturellement aussi de toutes les autres aides de la PAC, qui sera réformée avec notamment cette ambition, nous avons par ailleurs la conviction qu'il nous faut mener aujourd'hui une réflexion en profondeur sur la filière Blot pour son développement dans le cadre des états généraux de l'alimentation, comment expliquer que, face à une demande croissante des consommateurs pour le bio et après 5 ans d'aide à la conversion, les agriculteurs ne parviennent toujours pas à vendre leurs produits bio à un prix qui leur permettent d'en vivre, il s'agit là du défi à relever dans les prochaines années en amplifiant les efforts de tous pour que la croissance du marché bénéficie aux acteurs de l'agriculture biologique, ainsi qu'aux consommateurs, les agriculteurs bio ne sont, n'ont pas de raison d'être inquiets car nos objectifs pour le bio sont intacts, ils sont toujours de passer de 6 à 8 pourcent des des surfaces cultivées à la fin de la programmation de la programmation, voire plus car c'est possible et c'est le sens de notre ambition pour l'agriculture française, ils sont aussi d'atteindre en 2020, 2 50 pourcent de de produits bio de qualité et judiciaire qui court dans la restauration collective, je vous remercie. Merci, la parole est à notre collègue Henri Leroy pour le groupe, les républicains, vous avez la parole collègues. Monsieur le président. Là messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur 46 policiers ça gendarmes se sont donnés la mort depuis le début de l'année, la semaine dernière, 7 membres des forces de l'ordre se sont suicidés, un suicide par semaine depuis le début de l'année, un suicide par jour la semaine dernière, ces drames sont épouvantables et nos premières pensées vont aux familles de ses fonctionnaires, les forces de l'ordre font bien tous les jours leur travail, confrontés à la violence à une absence totale de respect de l'autorité, parfois même un rejet de ce que nous sommes les forces de l'or ne supportent plus le manque de soutien, le manque de moyens et le manque de considération, ils ne supportent plus d'être trop souvent narguer par ceux qui ne respectent pas la loi, insulté et menacé sur les réseaux sociaux, la recrudescence des suicides illustre dramatiquement un malaise très profond, c'est un épouvantable révélateur votre réponse Monsieur le Ministre, apparaît malheureusement bien convenu, la prévention des risques psychosociaux et votre priorité des psychologues Redden migration des cellules de veille déploiement de réseaux de référence, c'est important, mais il y a rien de nouveau là-dedans et c'est bien loin d'être suffisant, ne pensez-vous pas qu'il est temps pour redonner le moral à nos hommes d'appliquer la loi pénale sur notre territoire, qu'il est temps de sortir de l'angélisme qui nous mène aux polices de sécurité du quotidien et aux travaux d'intérêt général, il est temps de sortir de l'impunité dont bénéficie toute une partie des délinquants en France. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Henri le loi le roi, pardon, c'est avec une grande émotion que nous avons appris la semaine dernière que 6 fonctionnaires de police et 2 fonctionnaires de gendarmerie s'était donné la mort, je veux ici assurer leurs familles, leurs proches, leurs collègues de travail, de tout mon soutien de celui du gouvernement, de celui de l'ensemble de cette assemblée, il est toujours difficile d'expliquer de tels gestes dont les raisons sont multiples, dont les causes sont complexes, et si ce sont souvent des raisons intimes de maladie de vie personnelle qui explique le passage à l'acte, il est incontestable, monsieur le sénateur que la dureté des tâches de nos policiers et de nos gendarmes ne peut être éludée, eux qui doivent maintenir l'ordre public qui sont amenés à lutter contre le terrorisme qui traque Les criminels les délinquants sont en effet confrontés sans cesse à la violence à la désespérance et oui, cela peut amener à une tension et un stress extrême, c'est pourquoi, depuis plusieurs mois, de nombreuses actions ont été mises en oeuvre pour prévenir de tels actes, action pour le soutien psychologique aux agents le service dédié, doté de 80, psychologue pour la police et de 38 pour la la gendarmerie, sensibiliser les élèves policiers gendarmes dès la fin de leur scolarité, cellule de veille référant à l'accompagnement dans les commissariats et les Brigades mais pour réagir à cette situation, nous avons demandé dès dimanche au directeur général de la police nationale et au directeur général de la gendarmerie nationale, de mener une évaluation très précise de ces mesures, nous en tirerons toutes les conséquences, je voulais enfin vous dire que le ministre de l'Intérieur, va recevoir très rapidement, les syndicats de l'ensemble de la police sur ce sujet, je vous remercie. Oui, madame ministre votre réponse malheureusement montre également que votre logique et de traiter les conséquences plutôt que l'école, les forces de l'Ordre de retrouveront le moral lorsque la loi pénale sera appliquée partout sur notre territoire, lorsque les voyous faut conférant traités comme des délinquants et les policiers et les gendarmes respecter quand même le dehors. La parole est à notre collègue. Jacqueline Eustache-Brinio pour le groupe, les républicains. Le seul président, Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Jacques Mézard ministre la cohésion du territoire, des dizaines de Millau d'euros ont été consacrés aux quartiers depuis des décennies, lorsque l'on pose la question aux habitants sur ce qui a changé, ils vous répondent rien ou si peu, preuve des échecs successifs des politiques de la ville et politiques en faveur des quartiers ont consisté à saupoudrer beaucoup d'argent, une façon d'acheter la paix sociale aujourd'hui, après les annonces faites par le président de la République, quel désespoir pour les habitants de ces quartiers j'été maire jusqu'à ces jours derniers d'une commune, un quartier classé en petite de la ville, on expérience de terrain m'amène à penser que la question de l'avenir de lui et de nos quartiers en difficulté n'est pas tant une question de moyens qu'une question de volonté pour remettent la République au coeur des quartiers, il faut redonner du sens à l'autorité, il faut réhabiliter les valeurs de la République être intransigeant sur le respect et cela doit commencer dès le plus jeune âge, c'est la condition sine qua none pour y retrouver une qualité de vie et l'espoir d'y retrouver un emploi, le président de la République en annonçant pour les banlieues, des mesures dérogatoires et particulière, bien souvent déjà vu, comme par exemple les emplois francs ou le Neiman schème tombent dans le piège de la discrimination positive, non seulement, ces mesures ont peu de chances de porter leurs fruits mais ne croyez-vous pas, Monsieur le Ministre, Cannes constitue une entorse à l'égalité républicaine, ne croyez-vous pas que la discrimination positive en filigrane du discours du président la République est inspirée du modèle anglo-saxon, être contraire aux principes fondamentaux d'une République une et indivisible. On vous répondent : la parole au ministre de la cohésion des territoires Jacques Mézard la. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je crois que vous n'avez pas raison de dire que rien n'a été fait,

par des gouvernements successifs et que lorsque l'on va sur le terrain, il est nombres de quartiers où l'on peut constater que beaucoup de travail a été réalisé, donc quand vous dites quand vous dites : l'argent c'est une chose mais ça ne suffit pas, je peux vous suivre mais il faut de l'argent et d'ailleurs on nous reproche de ne pas en mettre suffisamment mais ce qu'il faut c'est une, c'est une volonté, là vous avez raison, mais là où je ne suis toujours pas d'accord avec vous, c'est qu'il s'agit pas de discrimination positive d'ailleurs, je vous renvoie à celui qui, le 1er a utilisé ces mots, hé bien cette discrimination, c'est pas de la discrimination positive que de rattraper que d'amener dans ces quartiers le droit commun de rétablir l'accès au service public, il y a des problèmes dans des territoires ruraux, mais il y en a aussi dans nombres de ces quartiers où il y a moins de postes qu'ailleurs, où il y a moins de commissariat qu'ailleurs et où, manifestement, nos concitoyens se trouve confrontée à à des difficultés d'accès au service public de mobilité et avec, il faut bien dire des situations exceptionnelles, quand vous avez des quartiers dans lesquels 60 pourcent de de la population est allophone, c'est-à-dire ne parlent pas le français, ou par l'une vingtaine de langues, nous sommes obligés de mettre en place et de travailler, ce que nous sommes en train de faire à des mesures pas spécifiques, des mesures permettant, je l'ai dit de ramener le droit commun de ramener la République dans ces quartiers et là où vous avez raison, c'est qu'il faut qu'il y avait de l'autorité, ce qu'a rappelé très fermement le président de la République et que dans ces quartiers la sécurité puisse régner comme ailleurs. Alors Monsieur Luis, moi je crois que nous aurons gagné et que la politique de la ville aura réussi lorsque la police pour aller travailler sans cercueil, c'est que les enseignants pourront et enseignants toute qui étude que les travailleurs sociaux accepteront d'y rester, bref que les habitants puissent vivre au quotidien dans un climat de paix sécurité auxquelles chacun d'entre nous a le droit. La parole est maintenant notre collègue Martin lévrier pour le groupe, la République en marche pour 2 minutes. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail, vendredi dernier, vous avez posé le 1er jalon de la professeure profonde réforme de l'apprentissage, promise par le candidat Emmanuel Macron nous le savons, la France compte aujourd'hui environ 7 pourcent de de jeunes apprentis tandis que notre voisin allemand frôle les 15 entreprises industrielles nous trouve plus de jeunes embauchés en apprentissage. Alors même que la rentrée est déjà loin, les centres de formation en apprentissage disposent encore de nombreuses offres qui ne parviennent pas à satisfaire situation paradoxale dans un pays dont 23 pourcent des des jeunes de moins de 25 ans sont aussi chômage. Malheureusement, la filière de l'apprentissage et méprisé par les familles par les jeunes, mais plus globalement par le système. C'est pourtant une voie de la réussite avec plus de 70 % pourcent pardon pardon d'emploi stable à l'issue. Nous ne pouvons que déplorer ce manque de considération pour l'apprentissage, qui facilite non seulement l'ascension professionnelle de nos jeunes, mais qui contribuent aussi à permettre à chacun de trouver sa voie, des jeunes qui ne trouvent pas leur équilibre dans le système scolaire s'épanouissent et réussissent grâce à l'apprentissage. Ce n'est donc pas un cursus de second rang, mais il y a plus une grande voix de réussite en complément de l'Éducation nationale avec des passerelles entre les 2 qu'il nous faut renforcer aujourd'hui le système d'apprentissage, de s'adapter aux aspirations des jeunes et aux besoins des entreprises. Il est un outil qui doit remettre en marche ascenseur social, une fois ce constat fait, je tiens à vous renouveler tout mon soutien à cette réforme qui doit faciliter insertion professionnelle des jeunes et qui transforme à notre économie et fera évoluer les mentalités, j'en viens à ma question, madame la ministre, dans le cadre des concertations collectif que vous avez initiée comment construire et vous un triptyque solide qui associera entreprise céphalées régions au service de ces jeunes en recherche d'emploi et de diplômes valorisant, je vous remercie. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Martin lévrier d'abord je vous remercie de votre question parce que je sais l'attachement de ne très nombreux sénateurs qui l'ont montré, dans le temps à la question : l'apprentissage, à commencer par son président et je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous, aujourd'hui, l'apprentissage, études de voies de réussite et pourtant elle est mal vu et décrié pourquoi je dis que c'est une voie de réussite parce que 70 pourcent des des apprentis trouvent un emploi et parce que de un sur 2 trouve un emploi dans l'entreprise où il a été embauché, pourtant il y a de très nombreux obstacles hop et c'est un paradoxe, vous l'avez souligné au moment où nous avons un 1000000 300 1000 jeunes en France qui sont ni en emploi ni à l'école ni à l'université, ni en apprentissage, et ça c'est un scandale, c'est un gâchis humain, c'est une perte d'opportunités économiques et c'est un risque pour notre cohésion sociale, donc oui l'apprentissage a besoin d'être

en présence aussi de Sophie Cluzel il y a qu'un pourcent d'handicapés parmi les apprentis et de leur rappeler celles avec les régions avec les partenaires sociaux avec les organismes consulaires, avec les CFA, les professionnels du secteur, nous pensons que nous ne pouvons pas faire juste une petite réforme car il y a beaucoup d'obstacles, un jeune ne sait pas comment trouver l'emploi 30 prises ensuite le CFA, il ne sait pas quels sont les débouchés s'il veut avoir un diplôme s'il pourra continuer, ce qui est le cas, ces diplômes jusqu'au niveau ingénieur l'entreprise, je vais pas faire la liste, maintenant vous connaissez les entreprises il y a de très très nombreux obstacles et course d'obstacles pour les entreprises, à commencer par le fait qu'on peut signer les contrats pendant 2 mois sur 12, et toute une série de règlements qui qui gênent et donc aujourd'hui oui cette concertation que j'ai confiée à Sylvie Brunet, qui préside la session, travail, emploi du 16 et pour nous très important et j'aurai le nerf de vous présenter au printemps prochain un projet de loi qui intégrera cette dimension de la transformation de l'apprentissage, c'est l'avenir de la jeunesse qui est en cause et je vous remercie d'avance de votre soutien. Merci, la parole est maintenant notre collègue Patrick Kanner. Pour le groupe socialiste et républicain, donner la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le 1er ministre j'étais à Tourcoing ce matin pour entendre le discours du président de la République sur la politique de la ville, un discours de conviction et je pense sincère dans ce domaine si complexe, si sensible, il n'y a pas d'ancien monde ou du Nouveau Monde, il y a crée les conditions d'un monde juste, où il n'y a pas de quartier perdu pour la République, Emmanuel Macron, a rappelé avec raison qu'il faut casser le cercle vicieux de l'assignation de fête à résidence et disons-le, des ghettos, il a raison d'affirmer que ce quartiers ne doivent pas s'habituer à la sécurité, il a raison, dénoncé le poids grandissant dans certains quartiers d'un Islam radical, sans angélisme mais aussi sans amalgame. Rappelant ses priorités, ses valeurs, Emmanuel Macron, n'a pas remis en cause l'action du gouvernement précédent, des gouvernements précédents qui avaient établi une nouvelle géographie prioritaire lancée avec succès l'ANRU de renforcer la loi SRU, créer les conseils citoyens établi dans chaque contrat de ville, un plan d'action contre l'arrêt de radicalisation mis en oeuvre la garantie jeunes rétabli les moyens au secteur associatif, que la droite avait largement amputé ou crée aussi le testing, aussi le testing, contre les discriminations, mais, mais Monsieur le 1er Ministre où est la cohérence entre la création expérimentale des emplois francs et la baisse drastique des emplois aidés, où est la cohérence entre l'annonce 2 milliards supplémentaires pour l'ANRU et le garrot financier imposée aux bailleurs sociaux sans qui il n'y a pas de rénovation urbaine, où est la cohérence entre le principe affiché d'une sanctuarisation des crédits de la politique de la ville et la suppression de 46 millions d'euros d'actions en plein été 2017 monsieur le 1er ministre il y a les preuves des mots, il y a l'épreuve des faits à une mobilisation nationale dans le respect des 5,5 millions d'habitants qui vivent dans ces 1500 quartiers mais surtout pas dans une logique comptable, ses habitants n'ont pas à se justifier de la part de leur appartenance à la République française.

je ne ferais ni le panégyrique, ni la critique de l'action que vous avez menées communiste de la ville, je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui où où nous venons de rendre globalement hommage à Georges Clémenceau, il est nécessaire d'avoir une vision qui dépasse ces critiques qui, que nous échangeons de manière très démocratique, vous avez raison de saluer les propos du président de la République, il a pris conscience, comme le 1er Ministre de la pas tard non écart dans sa campagne électorale, il avait beaucoup insisté sur ces questions de politique de la ville, hé bien il a très clairement exprimé la volonté de l'État d'avoir une forte politique pour aller de l'avant pour faire un plan de relance de cette politique de la ville, je ne sais pas, d'ailleurs, si le terme de la politique de la ville est aujourd'hui le plus approprié, il n'en reste pas moins que ce plan de relance que nous allons matin pour la fin du mois de février, nous le ferons en concertation, nous le ferons en co-construction tant avec les collectivités locales, qui sont eux en première ligne sur ces dossiers, qu'avec les associations, qu'avec les conseils citoyens parce que cette co-construction, elle est indispensable pour tenter de réussir cet enjeu qui est absolument aujourd'hui fondamental car nous sommes tous confrontés dans nos communes, dans nos départements, à ces difficultés, vous avez rappelé monsieur le ministre, qu'il y avait eu ce périmètre avec plus de 1500 quartiers prioritaires, je sais pas si c'était le bon découpage, on va pas le remettre en cause ce qu'il faut, ce sont des mesures fortes, des mesures interministériel porté par l'ensemble du gouvernement avec le concours, la concertation des collectivités et de tous ceux qui ont compris et qui savent aujourd'hui que c'est un enjeu national. Monsieur le 1er ministre dames et messieurs les Ministres, merci, je vous rappelle que nos prochaines questions d'actualité, auront lieu le jeudi 23 novembre retransmise sur Public Sénat et France 3 je vais suspende la séance ne soit reprise à 17 heures 50 pour la la suite de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, la séance est suspendue.

Donc, la séance est reprise. Richard collègues, j'ai le très grand plaisir au nom du Sénat tout entier de saluer la présence dans l'autre tribune officielle d'une délégation de députés du Burkina Faso. Conduite.

d'amitié France-Afrique de l'Ouest et membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, notre collègue a représenté le président du Sénat, aux Assises de la coopération décentralisée à Ouagadougou début octobre dernier où il a été reçu en audience Boehner Wendy Stanislas Sankara 1er vice-président de la représentation nationale les relations entre nos 2 assemblées sont anciennes et fructueuse, et nous sommes particulièrement sensibles à l'intérêt que la déviation porte à notre institution au nom du Sénat de la République, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue et je forme des voeux pour que son séjour en France soit profitable et contribuer à renforcer encore les Liens qui unissent nos 2 pays. L'ordre L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, je vous rappelle que la discussion générale est Close, nous passons à la discussion des articles du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale. En première partie, dispositions relatives à l'exercice 2016. Oui, pardon, j'ai pas entendu donc, oui, oui, oui. Monsieur a train. Le président, monsieur le ministre, chers collègues lors de chaque dépôt d'amendements, comme c'est le cas pour ce PLFSS la commission des finances, exerce un contrôle de l'article 40 de la Constitution, selon lequel je cite les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique depuis la mise en place de la LOLF en 2001 l'initiative parlementaire a déjà été fortement limité, d'autant plus avec la pratique établie du Sénat, refusant les demandes de rapports nous ne ret comprenons pas que des amendements soient déclarés il recevable alors que les parlementaires qui les déposent prévoit un gage financier sur le prix du tabac, les revenus des entreprises ou une cotisation additionnelle par exemple l'ainsi notre amendement demandant des cadres, la prime à la naissance avant l'accouchement, comme c'était d'ailleurs le cas avant 2015 a été refusée au motif qu'il y aurait un coût de trésorerie entre les 2 exercices comptables pour l'État de même notre amendement pour le remboursement de la procréation médicalement assistée pour tous les couper, les femmes seules, financée par la hausse d'une contribution sur les entreprises du tabac, a également été refusée il y a, je dois dire un véritable sentiment d'injustice et d'aléas sur le sort réservé aux amendements qui nécessiterait a minima une motivation claire de choc qui recevabilité prononcé par le président de la commission des finances, nous souhaiterions donc ce que le Sénat envisage une réflexion plus générale sur ce sujet pour garantir les droits du Parlement et de fait, l'équité entre les groupes politiques.

Pas d'explication de vote donc qui est pour. Il est content. Donc, l'article 1 est adopté. Ensuite, l'article 2.

Je vais mettre aux voix à l'ensemble de la première partie du projet de loi de financement de la situation sociale pour 2018 est-il des demandes d'explications de vote. La demande explication de vote qui est pour.

L'avis du gouvernement. Donc sur cet amendement de la commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour. Contre l'amendement adopté.

Oui merci Les personnes morales de droit public ou privé, ayant une activité dans le secteur concurrentiel, sont soumises à une contribution sociale de solidarité des sociétés dites, perdu, le chiffre d'affaires dépasse 19 millions d'euros depuis 2017, les très grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 1000000000 d'euros doivent s'acquitter en Suisse de la contribution additionnelle et contributions supplémentaires, la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, l'article 4 prévoit de supprimer cette contribution additionnelle mais aussi de rationaliser le c'est 3 S, entraînant une perte de recettes pour la sécurité sociale de 480 millions d'euros pour notre part nous sommes juste que les grandes entreprises participent au financement de la Sécurité sociale à la mesure de leurs moyens, cette nécessité d'autant plus forte que ce PLFSS va acter l'adossement du RSI au régime général, vous connaissez comme moi les inquiétudes des indépendants qui craignent à terme un alignement de leurs cotisations sociales sur celles du régime général, il ne serait pas juste non plus d'en faire supporter les causes, les conséquences aux salariés, la solidarité doit donc d'abord si exercer entre les entreprises et je reviendrai sur ce sujet à l'article 11 nous avions dénoncé d'ailleurs sous le quinquennat précédent la suppression programmée de la C3, sur 3 ans qui rompait ce principe de solidarité et nous n'avons pas changé d'avis pour ces raisons, nous proposons d'une part une réécriture de l'article 4 visant à maintenir la contribution additionnelle pour les très grandes entreprises et, d'autre part à remplacer le montant de 19 millions d'euros au-delà duquel les entreprises sont redevables de la C3 cesse par 760000 euros montant d'ailleurs pré-existants avant 2014. Sur cet amendement, l'avis de la commission. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre d'amendement rétablit la C4 est ce qui est une mesure de cavalerie consistant, sans augmenter les recettes, a imputé sur l'année 2017, une partie des recettes de ces 3 S 2018 supprime les abattements de là c'est 3 S adoptée dans le 4 dans le cadre du pacte de responsabilité, ce qui alourdit la fiscalité des entreprises de plus de 2 milliards d'euros, donc c'est un avis défavorable, vous le comprendrez. Avis du gouvernement. Défavorable. Donc je mets aux voix l'amendement 443 avec 2 avis défavorables de la commission du gouvernement qui est pour. il est content. L'amendement n'est pas adopté, je ensuite on voit l'article 4 article 4 qui est pour.

en effet la nouvelle commence conventions médicales conclues en 2000 16 ans se traduit par des augmentations importantes, des charges c'est évolution est en cohérence avec le virage ambulatoire annoncée mais il reste à s'assurer que ces dépenses nouvelles auront des effets restructurant réels organisateurs et limitant véritablement les hospitalisations évitables et ne se côtoient, non pas à de simples mais très coûteux effet revenu additionnel de ce point de vue, il manque encore un dispositif prudentiel sur la médecine de ville à la hauteur de la sur l'exécution de l'Ondam 2016 et très probablement en 2017 ans et défaut risque de dépassement en 2018, ce sont les raisons pour lesquelles l'amendement propose un rééquilibrage de l'article 6 et de l'article 54 pour un un partage plus équilibré de l'effort. Monsieur le président, comme le relève l'auteur de l'amendement, la régulation de l'Ondam ne peut porter que sur les crédits des établissements de santé, médico-sociaux car il n'existe pas de mécanisme pour la de réserve présidentielle pour la ville est une question importante, mais ne pourra malheureusement pas se régler de manière immédiate, à la faveur d'un amendement, vous comprendrez aisément, rectifiant les prévisions d'exécution de l'Ondam pour 2017, donc c'est une demande de retrait Monsieur chers collègues ou un avis défavorable. Un but du gouvernement. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, votre amendement consiste à transférer 100 millions d'euros, dépenses de l'Ondam du sous-abject il ville vers le sous-objectif, établissements de santé or compte tenu des dernières données disponibles, notamment sur l'évolution des dépenses de soins de ville toute modification porteraient atteinte en fait à la sincérité de la présentation du budget, nous sommes donc défavorable. Monsieur PELE va vous maintenez donc l'amendement est est maintenu pas l'explication de vote qui est pour l'amendement.

Qui est contre l'article 6 est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la 2ème partie du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018. Et ce qui des explications de vote, pas d'explication de vote qui est pour. Qui est contre. Donc c'est adopté. Donc la 3ème partie dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre financière la Secret social pour l'exercice. 2018. Dispositions relatives aux recettes au recouvrement et à la trésorerie donc article 7 donc j'ai 6 demande de de paroles sur l'article 7, monsieur Roland Courteau à la parole, pardon Monsieur Daudigny.

Oui, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, je souhaiterais rappeler que cet article met en oeuvre une des mesures phare du programme présidentiel annoncé de longue date, largement discuté tout au long de la campagne électorale, elle opère un allégement sans précédent des prélèvements sur les revenus d'activité, financée par l'augmentation de la CSG de 1,7 points, il s'agit d'une mesure globale de justice sociale pour répartir plus équitablement le financement, financement de la protection sociale en sollicitant les revenus du travail, les retraites, soumise au taux normal de CSG et les revenus du capital, certes, un effort de solidarité intergénérationnelle et demandé à 60 pourcent néanmoins cette hausse sera neutralisée pour 75 pourcent d'entre en compte, et eux, compte tenu de la suppression progressive de la taxe d'habitation, y compris pour une large partie de ce vivant en maison de retraite où en est les pensionnaires des Epad privés non lucratifs en bénéficieront directement grâce au dégrèvements dont bénéficient Néron les établissements avec la ferme volonté de soutenir cette mesure de justice sociale, l'heureuse, le groupe la République en marche, votera contre les amendements qui remettent en cause d'équilibres de l'article 7. Merci, la parole est maintenant Madame Laurence Cohen. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur et Madame la Ministre, mes chers collègues, l'une des intentions affichées du basculement des cotisations maladie et chômage sur l'ASF CSG de donner du pouvoir d'achat aux salariés du secteur public, on pourrait fort bien se contenter, pour aller plus vite, de majorer quelque peu le SMIC et d'inviter les branches professionnelles à ouvrir un nouveau tour de table de négociations salariales, mais nous le savons, le gouvernement s'y refuse et il privilégie donc cette fiction de la hausse du pouvoir d'achat que constituerait la disparition des 0,75 pourcent restants restants de cotisations maladie après le basculement de 98 et de la part salarié de la cotisation d'assurance-maladie, le problème c'est qu'il n'y a pas de hausse du pouvoir d'achat, pas seulement parce que les cotisations sociales sont un élément de la rémunération des salariés et que le fait de les réduire, revient donc à réduire la rémunération des salariés, on appelle cela : alléger le coût du travail, au motif que les salaires sont depuis quelques années, devenu un coup plus que la juste rémunération du travail accompli, ce n'est pas notre conviction, mais la réduction est double, si l'on peut dire, parce que le principe même de la Sécurité sociale, nous le connaissons toutes et tous ici et j'ai appelé dans mon intervention générale hier, c'est celui qui veut que, face aux événements de la vie, le salarié et sa famille ne reste pas sans ressources, qu'il s'agisse de la maladie de l'éducation des enfants, ou encore de l'interruption de l'activité, or, que voit-on dans ce PLFSS un basculement de la cotisation maladie résiduelle mais aussi un Ondam contraint à la moitié de son évolution naturel et cela pour les 5 années à venir, si l'on suit l'orientation de la loi de programmation des finances publiques pour le chômage, que doit-on penser au moment d'ailleurs où la négociation en cours sur les régimes de retraites complémentaires du secteur privé risque de s'achever avec un principe de mise en cause du niveau des pensions, je me permets de rappeler ici, avant de revenir sur toute autre considération que le système actuel d'indemnisation est plutôt défaillant et que le nombre de privés d'emploi, pris en charge par le régime Unédic et plutôt minoritaire, ce qui veut dire que toute indemnisation éventuelle des chômeurs se fait dans un contexte de rejouer, de ressources déjà insuffisant, nous sommes donc bien avec cet article 7 en face d'un véritable miroir aux Alouettes simples promesses électorales qui ne change rien au problème posé par le partage de la valeur ajoutée entre travail et capital, ni à celui de la répartition des gains de productivité, le salaire Direct ou non individuel ou socialisée n'est pas les ne nommer de l'emploi est non seulement injuste n'est inefficace et porte un coup très fort à notre système de protection sociale, c'est pourquoi nous voterons contre. Merci, la parole est à monsieur Dominique Vatrin non monsieur Vatrin passe son tour donc maintenant c'est Monsieur Maurice Antiste. Madame la Ministre, Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'article 7 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, acte le transfert des cotisations sociales vers la CSG ainsi pour compenser la suppression en plusieurs étapes des cotisations salariales maladie et chômage due par les salariés, le taux de CSG sera augmenté de 1,7 point pour tout le monde, actifs, retraités et fonctionnaires ce taux passera de 7,7 dès dès le 1er janvier 1900 2018 avec suppression des cotisations sociales en 2 fois le PLFSS annonce une baisse de 2,25 pourcent pour pour le 1er janvier puis le reliquat, le 1er octobre cela augmenterait certes le salaire de 132 euros par an en 2018 puis 263 euros en 2019 pour un un salarié payé au SMIC mais cela impliquerait également une hausse d'autant du revenu Net imposable avec des conséquences certaines sur les diverses prestations ou exonération dont peuvent bénéficier certains salariés, idem pour les autos entreprenant entrepreneur pardon et indépendant dont le taux de CSG de 7,7 pourcent et et passera à 9,2 concernant les retraités, le taux de CSG est actuellement à 6,6 pourcent et et passera à 8 3 dès le 1er janvier 2018, avec comme conséquence une baisse de leurs revenus, cela ne sera pas compensée par la suppression des cotisations sociales, ni par la revalorisation de 0,8 pourcent des des retraités au 1er octobre je tiens à ce titre, a rappelé que près de 80 pourcent des des retraités estiment que leur situation financière s'est déjà dégradée, les personnes dédommager au titre de la prestation de compensation du handicap seront pour le Pare lourdement impacté en effet, ces personnes sont assujettis à la CSG, mais ne paye pas de cotisation salariés cette mesure va spécifique spécifiquement concernant les dans familiaux qui vont voir ce prélèvement augmenter sans compensation, alors même que le dénouement sagement qu'ils perçoivent est déjà très faible, 75 pourcent du du SMIC horaire au maximum pour un nombre d'heures souvent très sous-évalué par rapport au temps qu'ils consacrent réellement à leurs proches, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, c'est d'ailleurs publiquement inquiété en ce sens, dans un communiqué en date du 17 octobre, c'est pourquoi j'ai déposé un certain nombre d'amendements sur cet article afin d'y introduire plus d'équité et de justice sociale. Si la parole est à monsieur Yves Daudigny. Merci Monsieur le Président Madame Monsieur le le ministre mais mais chers collègues. La CGI l'article 7 ouvre la discussion sur 3 sujets lorsqu'elle fut créée par Michel Rocard en 1991 la CGT avait pour objet d'élargir le périmètre de financement de la protection sociale et l'on pouvait parler de mesure de justice sociale avec l'élargissement à l'ensemble des revenus et en particulier aux revenus du Patrimoine et du capital,

l'augmentation de ces jets soit inférieur à élimination de cotisation mais 3ème sujet lorsque les bénéficiaires de revenus de remplacement ne sont pas compenser l'augmentation de CSG induit des transferts entre lesquels théorie de population, c'est le cas aujourd'hui, c'était pas le cas en 1997 ou sous le gouvernement Jospin l'augmentation de CSG des retraités fut entièrement compensée, nous n'approuvons pas, je l'ai dit hier en discussion générale ce transfert sur les retraités et nous proposons tout à l'heure un amendement pour supprimer cette disposition mais je voudrais Monsieur le Ministre du Budget profiter de votre présence pour vous poser une question des commentateurs évoquent la différence entre le Ghana les recettes provoquée par générée par l'augmentation de CSG dès le 1er janvier 2018 et les pertes de recettes dues à la diminution de cotisations quelquefois j'étais est évalué à 3 milliards ou même 3 milliards et demi alors Monsieur le Ministre est-ce que vous pourriez nous donner les chiffres précis de recettes nouvelles de CSG de perte de cotisations et éventuellement nous dire quelle est la destination de l'écart qui existe entre ses recettes et c'est entre ses recettes, d'une Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, juste quelques mots sur cet article 7 au nom de notre groupe des Républicains pour dire d'abord que nous nous saluons le transfert d'une partie du financement de notre modèle social du travail au fond de l'assiette du travail vers d'autres sources de financement donc cette CSG qui remplace des cotisations sociales nous paraît aller dans le bon sens on aurait prof préféré la TVA, c'est un vieux débat, mais Monsieur le Ministre, nous l'avions voté ensemble dans une majorité de 2012, un peu tardivement, hélas, cette fameuse TVA compétitivité qui devait remplacer une partie des charges qui pèsent sur le travail, on y voit que des avantages, puisque c'est la compétitivité c'est moines pour les salariés, à l'époque, c'est vrai que ça peut être une mesure de pouvoir d'achat, une mesure de compétitivité, c'est essentiellement sur les charges patronales et pas sur les charges salariales, toujours est-il que le groupe des Républicains, donc, se félicite de ce transfert, on prend un la baisse de, le, le, la, la CSG, on la prend quand même, même si on aurait préféré la TVA d'ailleurs je crois que il y a pas que dans notre groupe politique que certains d'ailleurs, on le verra dans les amendements auraient préféré aurait préféré le la TVA reste cette question des retraites des retraités qui ne sont pas compensés et retraités quand même modeste, hein, à partir de 1400 euros par mois, ça leur coûte quelque 300 euros par an, et eux ne sont pas compensés, notre, notre groupe, ce qui a d'ailleurs donné lieu à un amendement de la commission des des finances que j'ai présenté, qui a été adoptée en tout points de vue antique d'ailleurs avec celui du rapporteur général de la commission des affaires des Affaires sociales pour exonérer donc cette cette tranche de de près de 8 millions de personnes qui auraient cette somme annuelle à payer sans être sans être compensée, donc voilà ce que je voulais vous dire monsieur le ministre, s'agissant de la position du groupe D des républicains qui votera donc les amendements qui seront présentées par le rapporteur général, appuyé par le président de la commission et mes collègues et moi-même, de la de la commission des finances. Merci, la parole à Monsieur Daniel Chassain. Monsieur le président je suis président de la commission, Madame la Ministre, Monsieur le ministre, chers collègues, que l'article 7 c'est donc la suppression des cotisations sociales d'assurance-maladie et l'assurance chômage 3 pour 3,5 pourcent de de la rémunération brute des salariés pour un salarié au SMIC, ça fait un gain de 260 3 francs 3 euros et pour un salaire Net de 2000 euros ça fait près de 500 euros donc, là, cette mesure est équivalente pour les pour les indépendants, avec des baisses de cotisations famille accroissement de l'exonération des cotisations d'assurance-maladie et donc la compense pour les agents publics la compensation est prévu donc le financement se fait par une hausse de la CGT sur le revenu d'activité de remplacement, les revenus du Patrimoine des produits durant des produits de placement, les produits des jeux et des pensions de retraites : la hausse de la jet, ça vient d'être dit, ne concernera pas les retraités plutôt 35 ans qui paie, qui perçoivent moins de 1400 euros par mois, excluant ainsi 40 pourcent de de retraités, il y a encore des revenus les plus faibles, la suppression de la taxe d'habitation va compenser jusqu'à personne pour une personne seule qui gagne-t-elle sa 1000 euros par an donc l'objectif de cette mesure est bien de de redistribuer 7 milliards d'euros aux actifs alors nous pensons que les retraités doivent participer au financement de la Sécurité sociale, et aussi que les actifs c'est une participation selon nous interroger générationnel, je rappelle que la France a un déficit de 2200 milliards d'une dette de 2200 milliards et que la sécurité sociale est en déficit mais 1,7 points nous paraît trop élevé, nous souhaitons pour les retraités, limiter la CSG à 1 cela entraîne un 1000000000 2 de moins de recettes pour la sécurité sociale, contre 4 milliards 5 d'euros si l'exonération est totale, donc nous souhaitons effectivement arrêté les déficits et que la sécurité sociale soit en excédent éclat cadet soient remboursés en 2000 22 août 2023, mais nous pensons que 1,7 c'est un peu trop pour les retraités et nous pensons qu'il est possible de trouver un 1000000000 d'euros, ça n'est pas en difficulté du budget de la Sécurité sociale, donc, nous ferons un amendement en ce sens, merci. Si Madame Lienemann voulait intervenir vous avez la parole pour des raisons structurelles de principe et pour des raisons liées à l'état budgétaire qui nous est proposé, la première raison de principe est lié au fait que, je crois que notre financement d'asthme, de protection sociale mérite une clarification, autant on peut considérer que la santé et la question des allocations familiales pourrait s'apparenter à un droit universel garanti à toutes et à tous, autant il me paraît dangereux pour l'avenir de notre protection sociale, de considérer que la retraite comme le chômage, indemnisation chômage change de nature, c'est-à-dire devienne une aide au lieu d'être aujourd'hui une assurance collective, une forme de ce que certains appellent le salaire différé, c'est un vieux débat que nous avons depuis la Libération et ce n'est pas sans conséquences sur la manière de traiter les problèmes puisque quand vous êtes une aide, on finit par la conditionner à chaque débat budgétaire, Bercy trouve 1000 raisons pour vous expliquer qu'il faut soit la réduire, soit la et on finit par avoir des allocations chômage ou des retraites, qui dit qui fondent comme neige au soleil et on tue aussi une forme de solidarité nationale là donc je crois que c'est dangereux pour l'avenir, notamment le basculement des cotisations concernant le chômage, mais c'est d'autant plus vrai que nous le faisons sur la base d'une d'un transfert vers un impôt ou en tout cas un prélèvement injuste n'est pas un impôt progressif et d'ailleurs pour ma part, j'ai toujours plaidé pour la convergence j'ai impôt sur le revenu pour former un grand impôt structurant dans la fiscalité française, mais qui plus est, aujourd'hui, la part payée par le capital de la CSG est un peu près de 10 pourcent on le fait, et c'est là que la question du contexte pèse aussi à un moment où le capital va être exonérés très fortement de sa contribution aux efforts et aux besoins de la nation, à la fois par le l'impôt sur la solidarité qui a été, qui va être baissé et par le mécanisme de la flotte taxe alors c'est bien beau d'en appeler à la solidarité entre les retraités, fusse-t-il les plus aisés et les jeunes générations mais on tue complètement le débat entre la solidarité nécessaire entre le capital et le travail et de ce point de vue, il y a une disproportion qui me paraît tout à fait révélatrice d'un certain nombre de choix que je ne partage pas, je ne crois pas que dans ce pays il y a besoin à ce point d'alléger toute contribution du capital et donc faire de la CSG, un outil de redistribution dans ce cadre n'est plus ce qu'il avait été, il n'est pas progressive qui plus est, c'est donc un mauvais transfert qui nous est proposé. Merci monsieur Courteau vous étiez inscrit pas en a parole donc en 1er mais vous êtes passé en dernier. Merci président, oui, il y a bien quelque chose de vraiment nouveau et que jamais gouvernement n'avait osé faire c'est de baisser le pouvoir d'achat des pour améliorer celui des autres, là effectivement, on est vraiment dans l'entièrement nouveau dans l'inédit dans l'original, et même dans le révolutionnaire entre guillemets ainsi la CSG des retraités d'hôtel augmenter pour financer les allocations chômage auquel lui le retraité n'aura jamais droit partant de cette nouvelle conception de la cohésion sociale demain jusqu'à appliquer l'augmentation de la CSG aux allocations chômage aux d'amitié journalière autre chose qui est entièrement nouveau et inédit et original et les retraités ont été heureux de la c'est qu'avec une pension de retraite mensuelle de 1000 900 98 on on se situe dans la catégorie très envié des retraités dit aisés, c'est toujours bon à savoir ben voilà un PLFSS dure aux faibles avec l'augmentation de la CSG, panique, le projet de loi de finances sur lui paraît plutôt faible envers les nantis avec la flat taxe et l'allégement de l'ISF combiné et si chacune des 100 plus grandes fortunes françaises devraient bénéficier à moyenne d'un cadeau fiscal de l'ordre de grille de 5 millions d'Europe, tout cela est injuste la chronique et quant productif, nous sommes en effet comme en dans l'entièrement nouveau d'ailleurs que le FMI, qui n'est pas encore perdu gauchiste se permettre de rappeler que pour favoriser l'économie, mieux vaut prendre aux riches pour donner aux pauvres merci mérite mérite tout de même d'être rappelé et souligner ce que je voulais faire à propos de cette prise de parole sur article 7. merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la Ministre, peut-être répondront intervenant sur l'article 7 cas article très important de ce projet de loi de finances de Sécurité sociale et peut-être, si vous le permettez, ensuite un peu plus léger, hein, les explications des des amendements, même s'il y a beaucoup d'amendements qui concerne beaucoup de professions et beaucoup de questions auxquelles bien. Je répondrai à à à la majorité comme l'opposition parlementaire. D'abord, de quoi parle-t-on, parce que nous avons lu, même si, aujourd'hui, lors du débat, nous sommes éclairés par des discussions que nous avons la semaine nationale sur cette augmentation d'la 7 points de CSG de suppression de cotisations sociales, il y a 2 seuils qu'il faut retenir, et il faut les compléter, si j'ose dire, avec le projet de loi de finances. Notre vie parlementaire notre vie institutionnelle et c'est dommage d'ailleurs, le gouvernement s'est exprimé notamment par des propositions que j'ai pu faire pour la modernisation de la du bon débat parlementaire nous débattons du volet recettes de la loi de finances du PLF et puis des recettes du PLFSS dans 2 temps différents, et peut-être que cela nuit malgré tout au contrôle que les parlementaires pour le gouvernement, explication politique, le gouvernement a vis-à-vis de l'opinion, à travers les parlementaires mais en attendant d'être dans les pharmacies du Chanel qui nous permettraient de passer plus de temps sur le règlement un peu moins sur le budget, y un peu plus de temps sur les vols commun de recettes et des crédits budgétaires ou le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, nous sommes bien obligés de différencier PLFSS et P-F mais je voudrais quand même que l'on considère dans un temps du budget global de notre État que nous parlons à la fois la taxe d'habitation et en même temps de l'augmentation de la CSG et la suppression des cotisations, il y a 2 seuils à partir de 65 ans s'est mis à 1394 euros que va se provoquer cette augmentation de CSG pour les retraités contribuables français est en dessous de 65 ans, c'est 1289 parce que vous savez qu'à 65 ans, il y a un abattement et et c'est pour cela qu'il y a ce passage de 1989 à 1394 donc on ne sous 2394 euros de revenus pour une personne seule. Les retraités, il n'y a pas d'augmentation de CSG, je dirais même que pendant le minimum vieillesse, il y a une augmentation de 100 euros par mois, qui est prévue sur la chronique du gouvernement, c'est pour ça que lorsque j'entends dire que, évidemment, à 1395 euros, on n'est pas riche quand on est retraité, je suis tout à fait d'accord évidemment sur ses prises de paroles, mais je voudrais quand même remarquer que les petites retraites ce que nous avons à l'habitude de constater dans le territoire, particulièrement dans le mien, qui connaît un territoire industriels et d'agriculteurs. Retraité c'est parfois 600 700 800 euros et il existe en outre mer : des gens qui, notamment dans les territoires l'école connaissent une retraite à 250 à 300 euros il y a des retraites très basse, il y a des gens qui touchent des retraites en-dessous du seuil de pauvreté, la première des choses qu'il faut souligner, c'est que ce gouvernement augmente de façon sans précédent, le minimum vieillesse pour ceux qui effectivement sont concernés ceux qui sont entre le minimum vieillesse et 1394 euros connaissent une fiscalité la CSG a changé et ce qu'il soit plus de 1394 euros dès l'année prochaine, ils auront la neutralité de cette augmentation de CSG avec les discussions que nous aurons ce projet loi de finance de suppression d'un texte habitations pour 80 pourcent des des Français puisque jusqu'à 2500 euros nets de revenus pour une personne seule, donc, vraiment, nous prenons les cas les plus simples pour chacun puisse ici comprendre et il y a une suppression d'un tiers de la taille Xavi tation dès le projet OL finance de l'année prochaine, il y a donc une neutralité de fiscalité pour les contribuables, quand nous parlons d'augmentation de fiscalité pour les retraités, nous parlons donc dans le débat qui va nous amener à discuter pendant quelques soirées ensembles de personnes qui touche plus de 2500 euros nets par personne seule et il s'agit là après, d'un débat, savoir si on fait ou pas contribué ces personnes-là, plus 2500 euros nets de revenus ou non, le gouvernement met en place, non seulement la promesse du président de la République, mais aussi celle de la majorité élue à la semaine nationale et je crois que, ici ou là, il a été très largement suivie dans la campagne électorale : quel était le projet du gouvernement sur cette augmentation de CSG pour les personnes à plus de 2500 euros nets de revenus pour une personne seule et assume effectivement cette solidarité intra, générationnel,

d'abord répondre aux sénateurs Joyandet avec tous les métiers, estime que je lui porte que au moment de 2012 n'était pas parlementaire je n'ont pas pu voter, j'aurais bien voulu être encore plus jeunes sur les dans l'assemblée nationale je sais que vous prêtez beaucoup de vertus, monsieur le Ministre, je n'ai pas eu celle, quand même, je voudrais quand même souligner avec lui, il a eu l'honnêteté de le dire, que la TVA sociale est en fait une TVA emploi sans quoi leur c'est débat économique intéressant qui consistait à augmenter un point de TVA ou 2 points de TVA et à supprimer une partie des charges patronales évidemment ce débat sur la TVA sociale, la TVA emploi à TVA compétitivité c'est un débat qui traverse le pays depuis au moins 10 ans, qui a été mis en place à la fin de l'année du du quinquennat du président Sarkozy a annulé au début du quinquennat de Monsieur Hollande, mais entre-temps les temps où un petit peu changé qu'est-ce qui a changé, d'abord, c'est notre différence de groupes et de comptes de TVA de fiscalité avec l'Allemagne est notre 1er partenaire commercial au moment où François Fillon et Nicolas Sarkozy met en place la TVA sociale à la fin du quinquennat il n'y avait pas le taux de TVA que l'Allemagne et que la France, puisque je vous rappelle que sous le gouvernement précédent la TVA augmentée et il y a une différence qui est devenue plus importante avec nos collègues allemands, la 2ème, chose que je voudrais dire à Alain Joyandet, c'est que même dans le projet de François Fillon lors de débats présidentiels, il n'était plus question de supprimer de cotisations sociales salariales en nombres, puisqu'il s'agissait bien là encore de diminuer les charges patronales

le 1er c'est 0 charges sur les entreprises qui embauchent des personnes jusqu'à la catholique donc la suppression des charges patronales, souhaitée par la TVA, au sens où vous la défendez Monsieur le Ministre, elle existe dans le projet de loi de finances puisque nous allons voter ce que beaucoup de gens attendaient depuis très longtemps, la transformation du CICE en allégement général de charges, notamment pour les plus bas salaires, parce qu'on sait que c'est le problème d'embauche de principal pour nous pour pour pour nos chômeurs en France et donc j'allais dire que le 0 charge ou la baisse de charges massives va faire plus que 0 charge, vous en conviendrez avec moi à partir du 1er janvier 2009 est assuré est assurée par le projet de loi de finances de, de, de, de cette année. La 2ème chose, c'est que nous avons le souci et c'était pas le souci de ce que vous défendiez, et je vous reconnais bien là votre netteté, nous avons le souci d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés de ceux qui travaillent, partant d'un principe assez simple, que le travail doit payer et qui doit mieux payés parce que il est tout à fait évident de dire. Que leur ce que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est au SMIC et qui est une personne seule, par exemple, qui a élevé des enfants, et souvent dans des cadres ou malheureusement 1152 euros Net par mois, qui est le SMIC Net aujourd'hui, on n'a pas les moyens effectivement de faire vivre sa famille correctement et qu'il faut contribuer à ses d'augmentation de salaire comme on augmente les salaires qu'on augmente son pouvoir d'achat en baissant la fiscalité pour les ménages, c'est ce que nous faisons 10 milliards de baisse la fiscalité pour la taxe d'habitation qui touche des familles extrêmement modeste, vous le savez puisque, à partir de à peu près 11000 euros nets de revenus fiscal, on paye la taxe d'habitation dans notre pays, ça c'est du pouvoir d'achat très concrètement pour nos concitoyens, c'est une vie économique qui permettra, nous l'espérons, en tout cas les prémices que nous voyons sont positifs des dents dynamique de croissance et donc une augmentation de salaire par les entreprises, c'est tout l'intérêt des ordonnances travail la libération des énergies du président de la République et du 1er ministre mais c'est aussi la suppression des cotisations sociales de 3 avril 15. Que nous évoquons et qui verra une augmentation nette de pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés de France, quelles que soient leurs revenus, alors évidemment c'est assez différent d'une augmentation de TVA, plutôt que d'une augmentation de CSG parce que voyez, Monsieur le Ministre, la difficulté de l'augmentation de la TVA, c'est qu'elle aurait touché tout le monde, ils ne mouraient pas tous mais tous frappé, dit le poète, l'augmentation de la TVA de 2 points, qui était le projet de François Fillon, savez que dans la primaire, il y avait des candidats qui

On revient à 2500 euros nets, donc nous augmentons effectivement d'un virgule 7 points la CG pour ce compte 2500 euros nets et plus, mais l'augmentation de la TVA aurait touché tout le monde

viendrait à imaginer que les plus pauvres, nos concitoyens n'achète que les produits pour la cécité, il n'arrive pas d'acheter des véhicules de partir en congés ou d'avoir une vie que tout à chacun peut avoir donc l'augmentation de la TVA, c'est une mesure qui aurait touché tous les Français et c'est une augmentation généralisée de la fiscalité pour ceux qui n'auraient pas été tout à fait convaincu par cet argument de bon sens, je peux prendre 3 cas pratique, quelqu'un qui touche aujourd'hui 2500 euros nets, imaginons qu'il soit dans l'augmentation de ces gestes en compensation ta Xavi tation essayons d'être le plus sincère possible 2500 1 euros de

ils ont sensiblement la même augmentation de fiscalité, par ce que vous nous proposez monsieur le ministre, et est-ce que nous proposons, si on n'est pas contre 900 euros Net par mois, prenons un retraité de 900 euros Net par mois, il y a quelqu'un qui ne touche pas l'augmentation du mien, dit il y a, avion, encore une fois très sincère, pas des phénomènes, il ne touche pas l'augmentation de que nous prévoyons, effectivement, mais il n'a pas d'augmentation de fiscalité puisque l'augmentation de CSG, c'est à 1400 et là a les 2 points de TVA que vous proposez, Monsieur le Ministre, et il a donc si nous appliquons votre projet législatif si j'ose dire, par vos amendements il y aurait une augmentation de 150 euros de contributions fiscalité plus de 2 points de TVA alors qu'il n'a pas d'augmentation de fiscalité si les retraités en ce qui nous concerne, il y a même un gain de pouvoir d'achat si il travaille, donc l'augmentation de la TVA, si c'est un débat qui peut être intéressant, d'une part, la TVA sociale n'en est pas vraiment d'une puisqu'a touché charges patronales comblé par la transformation du CICE en baisse de charges et en plus elle est antisociale par définition par rapport à ce que nous proposons et qui effectivement une nouvelle solidarité je reviendrai ensuite sur une question très intéressante du modèle social et son financement, mais qui est une autre, une monsieur le ministre, vous n'avez pas évoqué mais c'est un tout, nous avons proposons quelque chose qui n'est plus dans le projet de la droite républicaine et personnellement je l'ai regretté, y compris dans le débat présidentiel, vous avez arrêté défendent les heures supplémentaires défiscalisées, ce n'était pas dans le projet présidentiel et j'ai même entendu le candidat à la présidentielle, qui représentait la droite des républicains, expliquant qu'il ne pouvait pas le faire parce que il y avait la fin du temps de travail et que ses maîtres du franc même tant qu'accélérateurs dans le projet de loi de finances, la progression des des finances publiques que le 1er ministre du président avec vous, a proposé la semaine dernière par ma voix, il y a la défiscalisation il y a même plus la des cotisations si j'ose dire, des heures supplémentaires qui sont prévues dans la, dans le projet de la finance que nous vous présentons et donc pour toutes ces raisons. Je crois, malheureusement Monsieur le ministre Joyandet que si votre argumentation est la bonne date de 10 ans et ce n'est pas une attaque personnelle que que de que de vous le dire : non, je me permettrais pas cher alors

et j'ai toujours pas défendu compris la primaire comme vous un candidat qui proposait pas d'augmentation de TVA. Et je me rappelle bien des meetings où il disait que ce qui est proposé était antisocial mais on a droit de changer d'avis, vous comme moi, la Cimade, la, la 2ème des choses, la 2ème des choses, c'était pour évoquer finalement. Une question que que pose le côté gauche de l'hémicycle et qui s'entend sur comment nous concevons la façon dont on finance le le la protection sociale, ce que propose le président de la République et de façon extrêmement claire dans sa campagne à et et je voudrais dire monsieur sénateur qui a évoqué le mot de révolutionnaire, mais effectivement, c'est à la fois l'originalité de la transformation, c'est de d'arrêter une société qui fonctionne et qui a bien fonctionné jusqu'à présent, mais une société qui fonctionne par par des cotisations et des statuts pour essayer d'un d'un système universel, il n'y a pas de secret dans la transformation de la protection sociale, que nous vous présentons et ça ne veut pas dire un seul instant que la sécurité sociale et même le le dialogue social autour de la sécurité sociale est oublié d'ailleurs mais avec madame la ministre de la Santé, charité, nous avons présenté le projet de loi de finances à Sécurité sociale à la commission des comptes de la Sécurité sociale, nous discutons avec les caisses, discutant évidemment avec les partenaires sociaux, ce que nous disons, c'est qu'effectivement, il faut que ce soit 2 points de vue universelle et non plus par statut qu'on doit financer une protection sociale et que, oui, nous sommes un gouvernement qui, qui, par la suppression de cotisation à une augmentation de pouvoir d'achat est à repenser notre modèle social, social et je pense que ce sera pour le bien être évidemment de nos concitoyens, monsieur le sénateur peut pose question finalement de. L'Avantage des recettes fiscales que nous pourrions avoir sur le mécanisme qui évoque le gouvernement, ce que nous faisons pour des raisons de finances publiques, mais aussi parce que nous souhaitons inscrire la suppression de la taxe d'habitation des projets Pas de finances cette à la fois un projet de loi finance de sécurité sociale et Édouard finance, qui respecte la trajectoire budgétaire et en même temps qu'met en place les réformes voulues par le gouvernement. Si je vais caricaturer mais j'attends, je dirais qu'au 1er janvier les Français, notamment les Français qui, qui travaillent, qui sont salariés vont connaître une baisse de 2 tiers de leurs cotisations et n'augmentation d'un tiers de leur pouvoir d'achat et en octobre puisque c'est fait en 2 temps : il faut connaître le tiers qui reste de cotisations à supprimer et 2 tiers d'augmentation du pouvoir d'achat, ce qui fait que pour quelqu'un qui est au SMIC, l'année prochaine, c'est une augmentation de pouvoir d'achat de 150 euros, puisque nous sommes en 2 temps et en année pleine 2019 d'à peu près 250 euros et vous me dites voilà, dans ce contexte-là, il y a donc des recettes fiscales de CG, qui ne sont pas répercuter si je comprends votre argument donc d'abord en année pleine, il n'y a pas de mécanisme qui fait du bien, si vous me permettez, votre question pose pour les prochaines à peu près le montant de gain pour l'État, en tout cas pour nos comptes publics est un peu plus de 3 milliards ça correspond exactement, vous remarquerez Monsieur le sénateur au montant de baisses fiscales que nous avons inscrit pour la baisse de la taxe d'habitation. Dire que nous avons fait le choix de pouvoir répercuter puisque son à peu près à 3 milliards par an dans la chronique jusqu'en 2020, ce que la baisse de la taxe habitation pour 80 pourcent des des Français, c'est à peu près 9 à 10 milliards d'euros, nous allons baisser la fiscalité en même temps de la taxe d'habitation et de la CSG et donc ça fait c'est ces 3 milliards, je voulais juste dire aussi que les chiffres que vous voyez et c'est pour ça que entre Sens, le débat qui consiste à dire vous augmenter la fiscalité pour les plus pauvres et pas pour les plus riches et totalement injuste puisque nous augmentons la fiscalité pour les personnes qui ont plus 2500 euros nets de revenus par an par personne et donc pas pour ceux qui sont en-dessous dessous par définition mais la CSG là aussi davantage de toucher le capital

que Michel Rocard l'avait évoqué ce qu'il ailleurs me permet, dire on va avoir ce débat s'est longuement dans l'hémicycle, même si certains pouvaient combattre le principe même de la CGT, que si je peux comprendre que le côté droit, l'hémicycle défendent la TVA c'est un débat sur est-ce que la TVA est plus juste ou pas que d'autres impôts, c'est un débat qui est très intéressant, j'ai plus de mal à comprendre et on l'a eu ce débat très longuement la semaine nationale, pourquoi le côté gauche j'ai viendrait à se remettre en cause un impôt qui par nature et redistributif et inventé par les sociaux-démocrates, si j'ose dire, quand même, Michel Rocard l'avait imaginé, je sais que cette vérité peut être un peu embêtant parce qu'elle mérite au moins il y a une cohérence moi je voudrais surtout dire que je n'ai pas entendu à part des dépenses nouvelles, ce qui n'est pas extrêmement original et je n'ai pas entendu de d'autres, d'autres propositions, à l'exception, celle de monsieur Jospin dès il a qu'a défendu d'alternative à notre modèle qui, je crois bien parce je le crois bien a été a été évoquée en tout cas je crois que ce que propose au gouvernement a le souci de la cohérence effectivement la transformation et ce n'est pas un petit article que l'article 7 vous avez bien raison c'est article tout-à-fait transformant et parmi les réformes de structures, le rapporteur général. Du budget n'est pas parmi nous ce soir, mais Monsieur Jordi représente la la commission des finances. Il a évoqué les réformes de structure et transformation de notre modèle au bout de quelques semaines, de quelques mois le gouvernement effectivement voilà Monsieur le le président je voudrais enfin terminé pour dire que il est extrêmement important que nous puissions liés dans nos débats, ce projet de loi de finance et la finance de la Sécurité sociale il y a plusieurs amendements qui concerne plusieurs statues plusieurs corps de métiers plusieurs domaines, dans laquelle les représentants de la nation, ont un intérêt particulier, je répondrai donc plus particulièrement à ses caisses.

444. Nous demandons ici la suppression de l'article 7 qui prévoit l'augmentation de la CSG de un virgule 7 mois rappelle que la CSG, la seconde recettes fiscales de l'État derrière la TVA, contrairement à ce qui est présenté par le gouvernement ce qui vient d'être dit, nous ne pensons pas qu'il s'agit du s'agisse d'une mesure favorable au pouvoir d'achat, bien au contraire, d'ailleurs, si telle était le cas, je pense qu'il aurait mieux valu tout simplement augmenter le SMIC dégeler le point d'indice des fonctionnaires et les pensions des retraités par exemple pense que féminisme qui aide pour la simplification simplification, vous devriez être d'accord avec cela plus particulièrement la hausse de la CSG ne sera pas compensée du tout pour 2 millions et demi de retraités modestes, vous avez rappelé les seuils d'imposition je les répète pas ici mais simplement Monsieur Bean et je dirais que nous ne considérons pas pour notre part que les retraités dont les pensions sont de leur de 1300 1400 euros seraient des riches, vous non plus vous l'avez dit, mais ni même ne feraient partie d'une mythique classe moyenne qu'il faudrait toujours taxés je trouve d'ailleurs scandaleux d'opposer ici des retraités qui gagnent 800 euros voire moins à des retraités qui en gagne 1300 euros, moi aussi j'habite Les de France et je trouve ce procédé tout-à-fait irrespectueux pour nous les vrais riches, et ça je crois que c'est l'important à dire, ce sont les 500 plus grandes fortunes de France qui ont gagné 600 milliards d'euros en 2016 auquel nous accorder encore 3 milliards d'euros de cadeaux, la suppression de l'ISF, sans parler du 1000000000 et demi accordé aussi avec la diminution des prélèvements sociaux et fiscaux, on y reviendra sur les dividendes au titre du prélèvement forfaitaire unique, enfin nous refusons cet article qui prévoit la suppression des cotisations en général et met à mal notre système de sécurité sociale et ses principes, à chacun selon ses besoins : chacun cotise selon ses moyens, non, monsieur le Ministre, vous ne pouvez pas vous dire du côté de je ne sais quelle révolution, vous travaillez d'ailleurs ici, à la remise en cause d'un système de solidarité conquis de haute lutte par les travailleurs, c'est la sécurité sociale et d'ailleurs, je voudrais vous le dire, différence entre cotisations et impôts, c'est que la cotisation des droits, des droits des prestations définies des droits à la participation des travailleurs à la projection co-gestion de cette part prise sur les profits des entreprises et je crois que c'est cela qui vous dérange-t-elle et le sens de votre politique. merci monsieur le président, Monsieur le ministre, comme c'est comme si habitude effectivement le 7, cet amendement vise la suppression de l'article 7 et comme c'est l'habitude depuis des décennies on exige toujours plus, toujours aux mêmes personnes à cette France qui travaille, qui se lève tôt et qui met un point d'honneur à gagner honnêtement ça vit et qui a pour objectif pour luxe diraient certains, d'acquérir un bien immobilier et ainsi mettre sa famille à l'abri des accidents de la vie des accidents sociaux des accidents économiques pour finir par transmettre ce bien à ses enfants, avec cette hausse de 22 pourcent de de la CSG pour les retraités, vous vous attaquez à ceux qui se sont levés tôt, ceux qui ont travaillé toute leur vie et pour certains d'entre eux, ceux qui ont mis leur vie en danger ceux qui ont combattu pour notre pays, pour son drapeau pour ses libertés, c'est ce que sont ces retraités, monsieur le Ministre, une catégorie de Français bien modeste en réalité qui ne fait que bénéficier du fruit d'une vie de labeur sa génération est aujourd'hui votre cible celles et ceux qui touchent 1000 3400 euros par mois votre mesure vise un gain de pouvoir d'achat pour les actifs, son efficacité est d'ores et déjà remis en cause par les travaux de notre commission on alourdit une fois de plus, l'imposition sur les revenus, vous aller toujours plus loin dans la fiscalité confiscatoire, une mesure insupportable pour des millions de retraités inacceptable pour nous, je ne résiste pas, enfin, Monsieur le Ministre, a rappelé le retournement de points de vue pour le pas dire le retournement de veste de notre ministre de l'Économie Monsieur le maire, qui préconisait hier, rappelez-vous, ce n'est pas si vieux dans son programme présidentiel, une baisse d'ampleur de la CSG dès le début du prochain quinquennat pour les revenus du travail et les pensions de retraite, mais également les fruits de l'épargne, il indiquait encore qu'elle bénéficierait à tous les Français, cette baisse importante est un gage de confiance dans le succès à venir des grandes réformes annoncées,

Merci donc sur ces 2 amendements, l'avis de la commission. C'est un avis évidemment défavorable puisque ces amendements sont en totale contradiction avec la position de la Commission, donc voilà, merci. Celui Ainsi, le président d'abord je voudrais donner un avis défavorable, 2 amendements, vous l'aurez compris d'abord dire à monsieur le sénateur du groupe communiste, je me suicide, 2 titres du groupe n'est pas tout à fait celui-là que je comprends son argumentation je ne partage pas, au nom du gouvernement et, effectivement, c'est un débat intéressant mais mais mais qui pourra effectivement se suivre sur un débat de société qui je crois a été tranché, si ce n'est pas réaction présidentielle au moins par l'action législative puisqu'il mais j'entends bien, et c'est pour ça que je vous réponse ce sénateur, je respecte tout à fait vos vos arguments et votre vision Dada société simplement ce n'est pas celui qui a été choisi par le par le gouvernement Monsieur Ravier d'abord, je crois que quand on on a une candidate à la présidentielle qui ne fait toute la campagne sur l'Euro, mais qui au lendemain dit que finalement on n'en sortira pas de l'Euro, je crois que dans ces conditions, la réversibilité des vestes peut être largement souligné je ne sais pas ses fabrications française en tout cas, mais elle est, elle est assez intéressante, la 2ème des choses Monsieur Ravier c'est j'ai du mal à comprendre votre argument qui se contredit du début à la fin que ce que dit au début vous taxer ceux qui, comme toujours, se lève tôt le matin, puis à la fin, vous terminez par dire qu'il faut souligner que, il y a ceux qui ont pu mettre de côté, de l'argent pour avoir de l'immobilier, c'est tout à fait leur droit, nous sommes quand même que dans le programme économique du Front national que que vous défendez encore, j'imagine, il y avait pas de suppression d'impôts sur les mobiles du tout puisque même Madame Le Pen était absolument opposés à toute suppression, y compris de de l'ISF. mettons ça de côté, justement, c'est ce que nous vous proposons ce Rallye, nous disons que la politique que nous menons, jusqu'à présent, c'est une politique qui malheureusement ne donne pas à ceux qui travaillent aux jeunes qui commencent leur travail. à ceux qui commencent à 1152 euros Net par mois, qui n'ont pas les moyens de ce pouvoir d'achat et que nous devons tous faire par plusieurs plans de la politique publique, c'est cas sur les ordonnances travail c'est le cas pour les heures supplémentaires, c'est le cas pour la suppression des cotisations, une augmentation de pouvoir d'achat et vous faites semblant et je voudrais aussi faire un miroir si j'ose dire, avec intervention monsieur le sénateur tout à l'heure, fait semblant de bloqués à 1400 euros de revenus, alors que le moment d'augmentation de fiscalité et qui est un moment assumer donc le gouvernement ne se cache pas et son petit doigt, c'est 2500 euros nets par personne, puisque vous avez d'un côté, le téléphone, ça c'était élèves qui seront votées en même temps et qui rentreront en janvier en même vigueur dans la même année et donc jusqu'à 2500 euros nets par personne, il n'y a pas d'augmentation de fiscalité alors oui au-dessus de 1500 euros Net par personne pour les retraités, il y a une augmentation fiscalité elle est assumée par le gouvernement, on demande effectivement une solidarité générationnelle, on a le roi tout à fait de la combattre et on peut tout à fait entendre qu'elles soient combattues. Simplement la démocratie, pour qu'elles soient respectueuses demande au moins qu'on puisse argumenter sur les vrais chiffres, que propose le gouvernement dans ses projets de finance des projets finances de sécurité sociale : avis défavorable, monsieur le président. Explications de vote Madame Lienemann. Lienemann. Entendu la réponse tout à l'heure de monsieur le Ministre, qui nous ramène à pourquoi ce système est injuste, qui est en train de nous expliquer qui vont payer la l'allégement de la taxe d'habitation par la CGT. Donc, en clair, vous êtes dans un mécanisme où vous allez, et après quand tous les collègues disent la CGT trop élevé, faut quand même s'interroger, vous êtes en train de mettre en place un système fiscal qui est un ambroglio dans lequel il y a une interférence entre ce qu'est le financement de la protection sociale, on peut avoir des désaccords, on peut tout ça est normal, mais tout est mélangé avec le reste de la fiscalité et notamment de la taxe d'habitation, moi je crois que ce système est dangereuse dans la durée, pourquoi, parce que pour, comme la base est injuste, la CGT retraités les actifs etc, on fait ce qu'on appelle en terme des niches fiscales puisqu'on fait des exemptions, alors on va faire de la compensation fonctionnaires on va plafonner pour les retraités de moins de 2500 plus 3 et puis au cours du temps, au cours du temps, comme tout ça ne va pas tenir et que l'on va pas avoir un système avec des fondamentaux juste tout ça va s'effriter, on va nous expliquer qu'on manque de ressources et on va baisser les prestations, voilà ce qui est enclenché, et donc moi je crois que ce système est d'autant plus dangereux, on pouvait attendent du président de la République qui prétend porter je construis prétend qu'il veut porter une vision d'avenir structurante pour un nouveau monde, mais on ne part pas sur un avenir la protection sociale avec du cafouillage fiscale telle qu'il est mis en oeuvre et je pense que derrière ce cafouillage en réalité ce fait se font des choix très injuste, j'ai parlé du capital mais parlons des salariés, des retraités, un salarié de 5000 euros par mois va avoir un allégement fiscal autour de 600 700 enfin, par un allégement fiscal va avoir 600 ou 700 euros mensuels de salaire supplémentaire mais le retrait des 2500

et moi je prends quelqu'un qui est à 5000 euros, du moins lui il va avoir 600 à 700 euros de salaire supplémentaire, car c'est en pourcentage, on peut parler du SMIC, ça c'est un vrai sujet autour du SMIC, mais pour les salaires élevés cela vont être favorisé par rapport aux retraités ayant les mêmes ressources, donc tout cela est injuste, globalement et scabreuse du point de vue de la durabilité de ce projet. merci Monsieur, monsieur Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Oui, mais merci Monsieur Président je voudrais moi aussi intervenir d'abord pour dire que je ne voterai évidemment pas pas ces amendements de suppression de de l'article 7 et donc que j'accepte que nous discutions écoutez continuons sur la CSG et la façon dont on pourrait adapter j'ai au budget du PLFSS mais je voudrais revenir sur 2 choses : d'abord sur ce qu'a dit fort justement monsieur Vatrin nous arrivons Monsieur, ministre à la suppression assurantielle du régime chômage ensuite de 2ème chose vous avez dans votre intervention, avec beaucoup d'éloquence au début de votre intervention et à la fin d'autres interventions dit 2 choses importantes, et je ne voudrais pas que ces 2 choses importantes échappent à l'ensemble de nos collègues, c'est déjà importante, c'est d'ailleurs la même chose, allez au début et à la fin, c'est de dire clairement que vous souhaitiez avec ce gouvernement, mettre en place un régime fiscal pour assurer l'assurance maladie pour assurer la famille pour assurer les différentes branches de de la sécurité sociale et vous avez aussi dit clairement que vous souhaitiez que les recettes

que ce qui était, budget de l'État qui a assuré la solidarité et ce qui était cotisations qui a assuré la formation assurantiel Dieppe FSS disparaissent dans le cas d'un d'un budget global contrôlé uniquement par Bercy, je crois que ce serait extrêmement dangereuse pour la santé, pour la famille pour la TMP et pour les retraites.

et je suis pas tout à fait certain qu'il y a des monstres, d'un côté les gentils de l'autre, parce que pour répondre à l'argument de Madame Lienemann, très franchement, vous pouvez distinguer dans l'hémicycle ce qui relève du PLFSS du PLF, vous pouvez distinguer de cotisation et ce qui relève de l'impôt, enfin, pour les Français. C'est la même poche c'est même budget et c'est même travaille, qui paye la fiscalité qui est payé, donc on peut avoir des débats l'pu finir. Mais il me semble d'ailleurs que dans la séparation qu'il peut y avoir entre le peuple et ses représentants, dont on faisons tout ce parti d'une manière ou d'une autre, il y a l'incompréhension et l'incohérence des politiques publiques qui ont été menées et il me semble que l'ancien gouvernement sous le président Hollande a payé cher un projet de loi de finances, qui était peut-être voilà qui ce qui est intéressant, qui était conforme aux engagements du président de la République précédent et puis après la finance de la Sécurité sociale, qui a augmenté très fortement et fiscalité pour pour nos concitoyens et on s'est étonné après avoir vu des applaudissements d'un côté et des oppositions de l'autre, que les Français en viennent à payer de la même poche donc attention que nos débats techniques ne cache pas la vérité de concitoyens qui effectivement à 1200 euros Net par mois, se demande bien comment ils vont boucler leur fin de mois effectivement besoin d'un système de santé protecteur d'un système familiale encourageant et d'une fiscalité qui n'est pas confiscatoire Madame Lienemann, vous dites la CGC en appoint juste. Si nous proposions augmentation intervient vous aussi la TVA, c'est un impôt injuste, ailleurs c'est la première ressources de l'État et puis j'imagine que si je parle de l'impôt sur le revenu, beaucoup d'entre vous trouverez c'est un impôt injuste. Et puis je pense que quand on va parler avec des habitations, c'est même l'argument du gouvernement et vous le savez bien, c'est aussi un apport juste doublement juste pour les collectivités locales, comme pour les particuliers, la taxe foncière dans les Verts locative dans les départs avec les sur, c'est aussi un impôt injuste dites-moi quel est un impôt juste d'ailleurs, je regrette que lorsque vous étiez aux responsabilités ayez pas mis en place par définition l'impôt est normal, c'est une contribution tout à fait nécessaire à la puissance publique et à l'intérêt général, mais enfin, ne faisons pas le débat de l'impôt injuste parce qu'il me semble que, pour le coup, et peut-être suis-je en minorité dans ce qui est ma culture politique, je trouve que c'est un des moins injuste des impôts qui existe, alors on peut avoir un argumentation comme vous le faites en prenant des cas extrêmes,

caché le fait qu'il transformer fondamentalement la façon dont il devait désormais financer la Sécurité sociale, la politique familiale, la fiscalité, de nos concitoyens, ça n'a jamais été caché, c'est le président de la République, il apparaît effectivement été là élu et je pense que si les résultats ont été cela pour continuer une politique qui a pu apporter à la France de grandes avancées, mais dans le monde a changé, tout à l'heure à monsieur le sénateur qui demandait très honnêtement, c'était quoi la différence fiscale de ressources pardon et je lui a répondu avec la plus grande honnêteté

et le roseau dans 2 étapes pour des raisons en même temps de responsabilité des finances publiques et le même débat la semaine dernière c'était tous les groupes politiques qui nous disait d'être responsables, on en faisait pas assez et on n'était pas assez dans la ligne proposée par la baisse des déficits, je constate que, on peut avoir des débats différents et on n'a pas forcément toujours la même esprit de responsabilité dont acte, mais Madame Lienemann je vous disais que nous avons fait le choix pour des trajectoires de finances publiques et de justice, de la fiscalité 2 blessés en même temps la taxe habitation la première année et d'avoir ce Rosso de CSG mais c'est 3 milliards en plus, il y a évidemment pas de lien de cause à effet, c'était une argumentation que j'avais pour monsieur sénateur et c'est pour une année à partir de 2019 les 3 milliards de baisses de fiscalité PFC 3 milliards dans lequel j'espère, c'est la dépense publique qui diminuera qui nous permettra de baisser cette fiscalité puis pareil pour après, donc, ne faites pas croire par une démonstration qui démontreraient que Socrate est un chat que a égal B que B égal, c'est donc à égale, c'est je pense que Molière a montré qu'à partir de ce moment-là, c'était sa fille qui est devenu.

D'abord sur une affirmation selon laquelle il y aurait un gain de pouvoir d'achat pour un grand nombre de nos concitoyens. C'est oublier un peu vite que, en même temps qu'on augmente la CSG, certes on diminue les cotisations sociales, mais aussi on diminue la page mais aussi les retraités l'an prochain au goût ne connaîtront pas d'augmentation parce que ce sera pour une année blanche, on augmente le forfait hospitalier, bref, il y a un certain nombre d'augmentations qui vont sérieusement amputé la les gains de pouvoir d'achat dont vous avez parlé il y a quelques instants, ce qui m'attendent par ailleurs aussi, c'est le fait que, avec la nouvelle CSG ou la l'augmentation, on va pas seulement en financer les dépenses sociales, mais ça va rentrer pour le supplément dans le budget de l'État si si j'ai bonne mémoire, mais ce sera à la louche. La CGT, avec l'augmentation de la 7 devrait rapporter 23 milliards supplémentaires, les exonérations de cotisations sociales, c'est 9 milliards et quelques et 4 milliards ça fait à peu près 14 milliards il reste pour l'État un Boni de 9 milliards d'euros, donc ça n'est pas simplement la préoccupation du pouvoir d'achat des salariés, c'est aussi l'intérêt de l'État, et si j'ai bien compris, vous nous indiquer que ça servira en partie à financer l'exonération de taxe d'habitation, ce qui signifie que pour ceux qui n'auront pas de compensation et je pense au 8 millions de retraités, c'est 8 millions de retraités vont financer la suppression d'une partie de la taxe d'habitation, puisque c'est les soldes, c'est les perdants et par conséquent c'est leur argent qui va servir à financer l'exonération de taxe habitation, ce qui est tout de même à la limite de l'indécence. Merci donc j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRC sur les amendements identiques 444 et 522 je rappelle que l'avis de la commission un défavorable et que avis du gouvernement est défavorable, donc il va être procédé au scrutin public.

Le scrutin est ouvert.

plus personne ne demande à voter, donc le scrutin est clos.

les résultats du scrutin sur les amendements identiques numéro 444 et 522 contre l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs groupes politique et notifié à la présidence, nombre de votants. 343. Nombre de suffrages exprimés 265 pour l'adoption 16 contre 249 donc les amendements ne sont pas adoptées.

alors que la hausse de la CGE et compensée pour les salariés, les personnes dédommager au type de la prestation de compensation du handicap seront impactés par l'augmentation du taux de un en effet, contrairement aux salariés, ces personnes sont assiduité à la CGT, mais ne paient pas de cotisations salariales, c'est plusieurs et spécifiquement touchés les aidants familiaux qui vont voir ce prélèvement augmenter sans compensation, alors même que les moi je manque il touche est déjà très faible, rappelons-le, 75 pourcent du du SMIC horaire maximum et pour un nombre d'heures souvent très est sous-évalué par rapport au temps qui est consacré, Helmand à leurs proches, alors qu'ils ne peuvent toucher comme maximum 1143 euros par mois pour un aidant parent isolé, ils s'offriront une pas de pouvoir d'achat supérieur à celle des retraités touchant au moins 2394 euros Net par mois, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, c'est d'ailleurs très justement publiquement inquiété de la perte de pouvoir d'achat pour ces familles comptant années dans la CSG acquittée par ces personnes ainsi passer de 8,2 à 9,9 ce qui est le taux le plus z'élevé qui est le taux applicable aussi aux revenus du Patrimoine après prélèvement de la CSG, le montant attribué pour une heure d'aide un proche percevant la PCH passer et notez bien le chiffre de 3,42 à 3 David 36 euros pour des raisons d'équité, il est ainsi proposé que les personnes dédommager type de la PCH sont exclus de la hausse de la CSG et en complément, Madame la Ministre, je pense qu'une façon générale, il serait fondamental de revoir de façon très pragmatique, la place et le statut des aidants familiaux, notamment pour l'accompagnement et l'évolution des parcours des personnes handicapées, merci beaucoup.

Monsieur le Président mais, messieurs, mesdames les ministres, alors que la hausse de la CSG est compensé. Pour les salariés, les personnes dédommager au titre de la prestation de compensation du handicap seront lourdement impacté par l'augmentation du taux de 1,7 points en effet, contrairement aux salariés, ces personnes sont assujettis à la CSG, mais ne paient pas de cotisations salariales. Je passe directement la conclusion puisque mon collègue le collègue précédent rigoureusement le même amendement pour des raisons d'équité, de justice sociale, il est ainsi proposé que la personne dédommager au type de la prestation de compensation du handicap la PCH soit exclus de la hausse de la CMU, quel est le sens cet amendement. Merci donc ensuite l'amendement 447 rectifier bis monsieur Dominique Vatrin. Oui, la prestation de compensation du handicap, qui permet aux personnes en situation de handicap et leurs familles, de compenser la perte de revenus les dents va elle être d'aussi victime de la hausse de la CSG, pourtant si cette hausse est compensée pour les salariés, les personnes dédommager de la PCH comme cela a été souligné seront lourdement impacté par l'augmentation du taux de 7, sans contrepartie puisque, contrairement aux salariés, ces personnes ne paient pas de cotisations salariales, cette mesure est d'autant plus injuste qu'elle frappera des personnes, des gens fragilité économique 75 du SMIC horaire au maximum lorsqu'ils ont dû arrêter de travailler, réduire leur temps de travail et pour honneur un nombre d'heures souvent très sous-évalué par rapport au temps qu'elle consacre également à leurs proches, le CNC c'est d'ailleurs publiquement inquiété dans un communiqué en date du 17 octobre de la perte nette de pouvoir d'achat pour ces familles comptant un et dans la CSG acquittée par ces personnes ainsi passer de 8,2 à 9,9 ce qui est le taux le plus z'élevé qui est le taux applicable aussi aux revenus du Patrimoine après prélèvement de la CSG, le montant attribué pour une heure d'aide un proche percevant le PS la PCH ainsi passer de 3,42 euros à 3,36 euros pour un montant maximum de 1152 euros par mois pour un et dans parent isolé, tout cela et d'ailleurs, je tiens à le souligner, contradictoire avec l'esprit même de la loi qui a créé dédommagement maximum correspondant à un SMIC Net et c'est ce qui est remis en cause ici, à l'inverse, pour des raisons d'équité, de justice sociale, nous proposons que les personnes dédommager petit de la PCH ouais, exclu de la hausse de la CSG. Merci, avis de la commission. Oui, Monsieur le Président, ça peut paraître paradoxal, mais la PCH revenus du Patrimoine. Ces bénéficiaires supporteront donc une augmentation de 1,7 point de la CSG, sans compensation par des baisses d'autres prélèvements si votre commission partage l'objectif poursuivi par cet amendement ne lui semble donc pas possible, ni souhaitable d'inscrire une telle dérogation dans le texte, en raison du risque de non-conformité à la constitution, que cela constitue le gouvernement s'est engagé devant l'Assemblée nationale, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, à apporter une solution à une réelle difficulté, elle pourrait prendre, vous l'avez dit, la forme d'une modification de la nature de la PCH ou de l'augmentation de ce montant, l'amendement va vous fournir, je n'en doute pas l'occasion de préciser vos intentions pour le moment c'est un avis défavorable sur cette amende. Merci monsieur le président, avec Madame la ministre de la Santé, d'essayer d'arrêter, nous avons donné effectivement Monsieur rapporteur général, il y a un signe d'ouverture important sur un sujet dont les sénateurs qui ont présenté des amendements ont raison

donc ce que je proposerais bien Monsieur rapporteur général et par vertueux envers les sénateurs, vous Monsieur Saint envoyée et pour les autres, c'est peut-être soit vouvoie. Tirez vos amendements en attendant l'idée qu'au second, lecture et vous le vérifierai nous souhaiterions transformer cela en du pas du pas du capital parce que votre amendement coûte 30 millions d'euros, alors que la transformation en revenu coûte à peu près 5 millions d'euros pour la même efficacité pour les personnes concernées notamment porteuses de 2 de et, sans doute, peut-être un peu mieux pour elle, puisque il y a un abattement pour ce qui concerne le revenu c'est pas du capital ou alors on adopte vos amendements et je donnerai un avis de sagesse pour montrer l'intérêt et l'engagement du du gouvernement, mais ce n'est pas vous prendre par surprise, que veut dire que la semaine nationale nous modifierons cela pour revenir vers un revenu qui je crois a les mêmes objectifs que voulait tout se poursuivre mais qui coûtera moins cher aux finances publiques, donc je crois que, devant la la foule qui qui qui qui s'esbaudir Monsieur le Président, je voudrais l'avis de sagesse, mais que chacun soit informé qu'en seconde lecture, les choses seront un peu modifié si la ministre est d'accord. Monsieur le ministre vous donner un avis de sagesse est-ce que vous levez le gage, puisque sur le moment, il y a une gueule. Peut-être que chacun peut faire un pas et que je monsieur même mais c'est sénateurs vont défend l'idée qu'ils vous retirer leurs amendements devant la confiance que inspire le gouvernement met sur prendra la parole, si jamais ce n'est pas le cas. Alors donc, ensuite, explications de vote Monsieur Savary. Oui, merci Monsieur le Président, la PCH une prestation de compensation du handicap, comme la pas se presse, question de compensation de l'indépendance polypes, personnes âgées dans cette PCH payer largement par les départements, pas suffisamment compensés par l'État, jeune, petite parenthèse, moi pour le département de la Manche, c'est 16 millions d'euros, la recette, c'est 5 millions d'euros annuels toujours identique, donc ça compense fermer la parenthèse est constitué cette prestation à la fois des techniques d'aide humaine ou d'un avis, donc c'est véritablement l'avancée par rapport à la loi 2005. Mais bien sûr effectivité avec contrôle derrière faut effectuer des heures, c'est contrôlé, on paye des heures avec une différenciation etc Les gens ont encore le choix me semble-t-il, avec la CTP, l'allocation compensatrice tierce personne qui existait déjà avant 2005 et qui était la compensation que donner sens infectivité c'était la un revenu véritablement l'ACTP tandis que la PCH et une compensation alors au jour joint ses revenus du Patrimoine pour les aidants. Sinon, ça peut pas être considéré comme une revenus du Patrimoine ou alors c'est une anomalie terrible, puisque c'est une compensation, ça peut être pour des améliorations du logement d'aide aussi à la voiture etc, dans le cas de cette compensation, donc je crois qu'il faut véritablement, revoir le dispositif parce que ce serait quand même aberrant

recettes par le biais des sièges supplémentaires, madame la présidente, ce président ne contredira pas et ce serait quand même assez sidérant que ce soit encore l'État qui arrive à se faire là-dessus une gratte, je dirais, excusez-moi l'expression, par rapport au coût quand même devenant insupportable pour certains départements et je pense que les coûts parce que c'est bien sûr pour les personnes handicapées, quelque chose de tout à fait important pour lequel il faut aller et voyez-vous pas suffisamment de personnes ont choisi la PCH par rapport à l'ACTP, et je crains que si on n'accepte pas l'amendement, hé ben on arrive encore dans quelques années avoir que cette PCH n'a pas réussi entièrement son objet.

dans cet esprit de l'amendement qui a été de poser pour autant, pour reprendre l'argument que faisait Monsieur rapporteur général le, le fait de d'adopter cette cet amendement poserait une un problème d'ordre constitutionnel revaloriser la PCH en inscrivant en 2ème lecture dans la loi de finance, comme l'a suggéré, Monsieur le ministre à l'Assemblée nationale le 25 paraît tout à fait correct et nous garantirons de cette façon, aussi bien l'effectivité de la réforme que la priorité accordée au handicap par le gouvernement.

mais quoi qu'il en soit, je souhaite conserver l'amendement en ayant vos explications parce que je crois que pour le monde du handicap, c'est un signe important mais bien entendu nous ferons en sorte de regarder de très près les discussions à l'asthme nationale et je crois d'une façon générale, départ beaucoup de sénateurs, ici présent, il faut qu'on veut de façon globale le dispositif en tous les cas, sachez que nous le maintenons mais dans un esprit vente de de pouvoir travailler sur cette évolution. Donc l'explication de vote Monsieur Chassaing. Ce ministre effectivement la PCH considéré comme Patrimoine ça ça ça m'était complètement inconnu, donc il s'agit donc d'une d'une injustice, donc il faut sûrement revoir ce dispositif, parce que ça doit être considéré effectivement comme comme un revenu. Merci donc Monsieur train j'ai pas. Oui, pour dire aussi que nous maintiendrons cette un un amendement car nous pensons que le le vote qui devrait s'exprimer ici sera un encouragement à régler cette situation un signal fort envoyé aussi au monde du handicap qui attend effectivement ceci.

Monsieur le président, moi j'ai écouté, Monsieur le Ministre, nous dire voter l'amendement, même s'il est pas très constitutionnels, mais à l'Assemblée, nous essaierons de trouver la solution. j'ai, j'écoute, je suis pas mandatés par la Commission, elle a dit la commission s'était défavorable pour les raisons que je viens d'évoquer, donc j'ai quand même, j'ai plutôt le sentiment que la bonne volonté de Monsieur le Ministre de doit pas être découragé donc je proposerais bien volontiers à titre personnel de voter cet amendement dans cet espoir que Les handicapés que les personnes qui ont un handicap évidemment peuvent nourrir. Très bien, donc plus d'explication de vote j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains sur les amendements identiques 168 402 et 447. puisqu'il émet un avis, la commission est devenu favorable et l'avis du gouvernement et d'une sagesse bienveillante puisque le gage serait levé.

Le scrutin est ouvert.

Oui, plus personne ne demande à voter, donc le scrutin est clos. Eh

bien, voici le résultat donc du scrutin sur les amendements identiques numéro 168 rectifier bis 412 rectifier 447 rectifier bis continue d'ensemble, délégation de vote accordé par les sénateurs ou politique et à la présidence.

Voilà donc sur ce vote mais unanimes : je vais suspend la séance, elle sera reprise à 21 heures 30 pour la la suite de l'examen de ce texte, la séance est suspendue, monsieur, attendez avant de suspendre l'ASEAN je reviens. 15 secondes en arrière, le monsieur le président de la commission des affaires sociales, Alain Milon. Donc Monsieur Président, c'est juste pour dire au au sénateur, membre de la commission d'affaires sociales que nous avons réunion maintenant pour continuer de regarder les amendements.